La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 10 février 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. ... Le procès-verbal est adopté. Par lettre en date du 15 février 2021, le Gouvernement demande que la suite de l'examen de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification soit inscrite à l'ordre du jour du jeudi 18 février, matin, et, éventuellement, à la suite des textes préalablement inscrits de l'après-midi et du soir. En conséquence, l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux et sur le projet de loi relatif au code de la justice pénale des mineurs est avancé à ce soir. Acte est donné de ces demandes. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage

Monsieur le président, madame la rapporteure, chère Elsa Schalck, mesdames, messieurs les sénateurs, le dopage et, plus largement, les conduites dopantes ou addictives sont un fléau en ce qu'ils menacent l'intégrité de nos compétitions sportives comme la santé de nos sportifs, professionnels et amateurs. Au-delà, ils faussent la performance, pénalisent les athlètes propres et attaquent fondamentalement l'esprit de loyauté et d'équité, qui fonde pourtant l'essence même des compétitions sportives. Je salue à cet égard la décision du tribunal arbitral du sport du 17 décembre 2020, qui, grâce aux investigations menées par l'Agence mondiale antidopage (AMA) durant presque quatre a reconnu la responsabilité des autorités russes dans la dissimulation organisée d'échantillons positifs et un programme centralisé de dopage entre 2011 et 2015. La crédibilité de nos compétitions et la loyauté entre sportifs passent ainsi par des sanctions exemplaires lorsque les compétitions sont faussées. J'en suis intimement convaincue, une politique efficace de prévention du dopage est une politique qui est l'affaire de tous

corps médical, communauté scientifique, médias, sponsors, mais aussi l'ensemble du public amateur de spectacles sportifs. Aussi, dès mon arrivée au ministère des sports, en septembre 2018, j'ai tenu à placer les enjeux d'éthique au coeur de mes priorités. Je considère en effet que le ministère des sports doit s'investir prioritairement dans les politiques publiques liées à la protection des pratiquants, qu'il s'agisse du sport de haut niveau ou du sport amateur. Jean-Michel Blanquer et moi-même poursuivons une politique volontariste de lutte contre le dopage et toutes les formes de conduites addictives. Cette politique associe l'ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles Ensemble, nous développons des programmes de formation et de sensibilisation des sportifs et de leur entourage ; nous accompagnons les fédérations et les établissements du ministère dans leur campagne de prévention et l'élaboration de leur stratégie nous donnons les moyens humains et financiers nécessaires à une lutte efficace contre le dopage. L'efficience de notre politique passe en effet nécessairement par les actions concrètes que nous menons. Durant ma carrière de nageuse de haut niveau, j'ai profondément manqué d'informations sur les produits à risque et la lutte contre le dopage. Avec Witold Banka, le président de l'Agence mondiale antidopage, lui aussi ancien sportif, je partage la même détermination à former et impliquer les sportifs dans la préservation des valeurs de notre sport. Le plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes 2020-2024 et le guide d'accompagnement à destination des fédérations sportives illustrent ainsi l'engagement des pouvoirs publics français pour renforcer une culture commune de prévention et de vigilance, à tous les niveaux de l'organisation sportive. Je présiderai d'ailleurs un comité de pilotage de ce plan national le 23 février prochain, pour faire un point d'étape avec tous les acteurs concernés. L'engagement de l'État en faveur de la lutte contre le dopage est bien sûr aussi financier en 2021, ce sont près de 12 millions d'euros que notre gouvernement investit en soutien des opérateurs de la lutte contre le dopage. La contribution annuelle de la France au fonctionnement de l'AMA s'établit, ainsi, à plus d'un million d'euros. Par ailleurs, la dotation attribuée par l'État à l'Agence française de lutte contre le dopage atteint près près de 11 millions d'euros, pour permettre notamment des recrutements complémentaires ainsi qu'une augmentation du volume des contrôles, qui passeront ainsi de 7 000 à 10 000 en 2021. Notre ambition s'inscrit dans la perspective de l'accueil à Paris des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Cet événement planétaire doit nous permettre de changer la place du sport dans notre société, de l'inscrire durablement dans le quotidien de tous et, bien sûr, d'en faire le véhicule central d'un sport propre, loyal et digne. J'en viens plus précisément au sujet pour lequel nous sommes réunis cet après-midi, à savoir la transposition des nouvelles dispositions du code mondial antidopage dans notre droit français. Ce code, vous le savez, n'a pas de force contraignante directe à l'égard des États.

Permettez-moi de rappeler brièvement la chronologie qui me conduit devant vous aujourd'hui, dans le cadre d'une procédure accélérée. La version 2021 du code mondial antidopage a été adoptée en novembre 2019 en Pologne. Dès le 19 février 2020, j'avais déposé un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale, dont l'examen n'a malheureusement pas pu s'inscrire dans l'agenda parlementaire compte tenu des urgences liées à la pandémie. Le 7 décembre dernier, les députés ont adopté à l'unanimité l'article unique du présent projet de loi, qui vise à habiliter le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage. Je l'avais dit à l'Assemblée nationale, j'aurais souhaité pouvoir offrir, pour la première fois, un débat de fond à la représentation parlementaire sur les prochaines dispositions législatives du code du sport en matière de dopage. Malheureusement, la crise sanitaire a bouleversé notre calendrier législatif. Je suis donc contrainte de procéder, comme les précédents gouvernements, par voie d'ordonnance, avec la confiance du Parlement. Dans le cadre des travaux parlementaires menés avec Mme la rapporteure et les membres de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, j'ai écouté les préoccupations exprimées et tenté de lever les inquiétudes. Devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite réitérer les engagements pris par le Gouvernement. D'abord, concernant les pouvoirs d'enquête qui seront confiés à l'AFLD par la future ordonnance, le travail conjoint mené avec l'AFLD nous a permis de considérablement renforcer les prérogatives dont disposera l'Agence pour mener le plus efficacement possible une lutte antidopage complémentaire des procédures judiciaires pouvant être parallèlement engagées. Comme aucune autre organisation antidopage nationale, les enquêteurs de l'AFLD pourront ainsi user d'une identité d'emprunt sur internet, accéder aux locaux professionnels et sportifs, se faire communiquer tout document utile ou encore convoquer et entendre toute personne de l'entourage d'un sportif en amont d'une procédure disciplinaire. Le travail de rédaction de l'ordonnance a été long et minutieux, car, comme vous, je suis profondément attachée à préserver les libertés individuelles et la présomption d'innocence. Quant au transfert, en janvier 2022, du laboratoire d'analyse au sein de l'UFR (unité de formation c'est une chance immense pour notre lutte antidopage d'intégrer ce campus récemment reconnu « initiative d'excellence » par un jury international. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, le ministère a accéléré la mise en oeuvre d'une collaboration rapprochée avec l'université. Vous nous avez permis de faire progresser ce projet, afin d'en faire un laboratoire d'excellence ; je tiens à vous en remercier. Désormais, un comité de pilotage se réunira tous les mois pour mettre en oeuvre efficacement cette réforme et traiter de tous les sujets de façon positive. Ce comité a vocation à élaborer le futur modèle économique du laboratoire, au travers de trois perspectives qui l'assureront de son rayonnement national et international : son fonctionnement courant, ses capacités d'investissement pérennes et la gestion de ses fonctions support. Dès 2022, le ministère chargé des sports apportera à l'université des ressources à la hauteur de nos ambitions communes, pour la qualité des analyses, les investissements en matériels ainsi que les travaux de recherche. Une convention pluriannuelle liant l'État à l'université apportera toutes les garanties nécessaires. Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que, pour vous, le sujet de la lutte contre le dopage ne souffre aucune polémique partisane. Très bien ! Le texte de l'ordonnance, que j'ai tenu à transmettre en toute transparence à la commission présidée par M. Laurent Lafon, recueille l'accord de l'AFLD et celui de l'AMA. J'envisage d'en saisir le Conseil d'État dans les tout prochains jours, pour être en mesure de présenter l'ordonnance définitive en conseil des ministres avant la fin du mois de mars. Ainsi, nous pourrions, ensemble, avoir finalisé la transposition législative complète avant la date limite fixée par l'Agence mondiale au 12 avril prochain. Je tenais, pour finir, à saluer la grande qualité des travaux de Mme la rapporteure et les échanges constructifs que nous avons pu avoir. Très bien ! Je tiens également à remercier les équipes du ministère des sports et de l'AFLD pour leur travail, si précieux dans la rédaction du texte de l'ordonnance, qui se prolonge d'ores et déjà avec la mise à jour de la partie réglementaire du code du sport. Mesdames, messieurs les sénateurs, je compte sur vous pour nous permettre d'adopter ce texte dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. La parole est à Mme

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi d'habilitation que nous examinons aujourd'hui est très technique, puisqu'il s'agit de permettre au Gouvernement, par voie d'ordonnance, de modifier plusieurs dizaines d'articles du code du sport pour les rendre conformes aux prescriptions du nouveau code mondial antidopage, adopté à l'automne 2019 dans le cadre d'une conférence internationale organisée par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Si les dispositions concernées par le projet de loi sont effectivement complexes, ses principes et ses objectifs sont au contraire très simples : ils visent tout simplement à renforcer l'éthique du sport. Les questions qui se posent sont fondamentales comment garantir l'équité des chances entre les sportifs ? Comment s'assurer que les comportements irréguliers seront identifiés, jugés et sanctionnés ? Comment préserver la santé des sportifs, lutter contre les tentations et dissuader les tentateurs ? Comment, enfin, créer une vraie culture de la prévention, grâce à la formation et l'information des sportifs et de leurs encadrants ? Madame la ministre, nous partageons complètement votre souhait que le nouveau code mondial antidopage, qui comprend de nombreuses dispositions utiles pour rendre l'arsenal antidopage plus efficace, puisse être adopté au plus vite. Le dopage est un véritable fléau qui doit être combattu, car il nuit aux valeurs mêmes que le sport véhicule. Nous avons par ailleurs un devoir d'exemplarité dans la perspective des grandes compétitions que nous allons accueillir, qu'il s'agisse de la coupe du monde de rugby en 2023 ou des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Nous sommes donc résolument favorables aux dispositions prévues par ce nouveau code mondial antidopage, qui marque un changement de nature de la lutte antidopage, au travers de la mise en place d'une politique publique plus collégiale privilégiant la prévention grâce à l'information et à la formation.

Vous nous l'accorderez, le Sénat n'est pas responsable du fait que nous n'examinions qu'aujourd'hui, le 16 février 2021, ce projet de loi qui aurait dû être adopté voilà plusieurs mois, pour permettre au nouveau code d'entrer en vigueur au 1 janvier 2021. Dans ces conditions, quel est le rôle du Sénat ? Devons-nous adopter ce texte sans poser de questions, pour vous permettre de rattraper un peu le retard accumulé depuis plus d'un an ? Bien évidemment, le Sénat ne pouvait faire l'économie d'un travail de fond sur le contenu du code mondial antidopage et les problèmes engendrés par sa mise en oeuvre. Nous avons donc longuement auditionné l'ensemble des acteurs au mois de janvier, afin de nous faire notre propre opinion. Comme vous le savez, ces auditions nous ont été précieuses pour identifier au moins deux sujets de préoccupation, qui n'ont pas permis à la commission d'adopter, voilà quinze jours, Je reviendrai sur ces deux points clés. À ce stade de nos échanges, je souhaite vraiment que les enjeux du débat d'aujourd'hui soient parfaitement clairs pour chacun d'entre nous. Nous sommes conscients de l'intérêt qu'il y a à ce que le Sénat apporte son soutien à ce texte. Nous souhaitons tous une plus grande efficacité dans la lutte contre le dopage et le nouveau volet relatif à la prévention nous semble très prometteur pour renforcer l'éthique du sport. Nous avons bien mesuré, par ailleurs, la contrainte de la date du 12 avril 2021, qui marque le terme du délai donné par l'AMA à la France pour se mettre en conformité. Mais le respect de ce délai ne peut avoir pour effet de nous priver des réponses que nous attendons sur les points qui font encore débat, d'autant que la date du 12 avril prochain constitue seulement une étape de la procédure de mise en conformité de l'AMA. Il n'existe donc aucune épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui justifierait de nous priver d'un débat. Notre débat d'aujourd'hui est utile. Je souhaite d'ailleurs saluer, madame la ministre, la qualité de nos échanges. Vous-même et l'ensemble de vos collaborateurs avez été à l'écoute de nos interrogations, et je peux d'ores et déjà indiquer que vous avez commencé à apporter des réponses très positives à nos demandes d'éclaircissement. Il est donc important, pour tous les acteurs du monde du sport, que vous puissiez cet après-midi nous confirmer ces avancées, mais aussi nous rassurer sur les quelques points qui demeurent en suspens, comme le confirment d'ailleurs les de tenir. Quels sont les sujets sur lesquels nous souhaitons vous entendre ? Ils sont au nombre de deux. Le premier sujet concerne les pouvoirs d'enquête administrative de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD. Ces pouvoirs sont aujourd'hui notoirement insuffisants pour lui permettre de remonter les filières et confondre tous les intervenants. L'AFLD demande depuis des années à obtenir des pouvoirs similaires à ceux dont disposent d'autres autorités indépendantes comme l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Or nous savons que le travail gouvernemental n'avait pas permis, jusqu'à récemment, d'aboutir sur la question de ces pouvoirs d'enquête. Notre commission s'est donc engagée pour demander que l'AFLD dispose au moins de deux types de pouvoir d'enquête administrative : un pouvoir de convocation assorti d'un pouvoir de sanction pour les contrevenants et un droit à recourir à recourir à des identités d'emprunt, notamment pour réaliser des « coups d'achat ». Je précise que l'AMF bénéficie de ces deux compétences. Nous le savons, vous vous êtes saisie ces derniers jours de ce dossier, qui a bien avancé. C'est pourquoi nous vous serions reconnaissants de nous préciser quels seront précisément les pouvoirs d'enquête de l'AFLD définis par l'ordonnance. Le second sujet est également important à nos yeux puisqu'il concerne le laboratoire antidopage, qui doit quitter le giron de l'AFLD pour rejoindre la faculté de pharmacie de l'université Paris-Saclay. Nous avons découvert, en auditionnant la présidente de cette université, que, à quelques mois du rattachement, elle ne disposait d'aucune indication sur le futur modèle économique de ce laboratoire, sur son budget prévisionnel et sur la prise en charge de sa masse salariale, alors même que le déménagement aura pour conséquence de priver le laboratoire des fonctions support que lui prodiguait jusqu'alors l'AFLD. Nous avons également été surpris d'apprendre que l'université n'avait jusqu'à présent reçu aucun accompagnement pour organiser ce rattachement. Nous savons que, là encore, vos services se sont saisis du dossier et ont décidé de mettre en place le comité de pilotage, qui n'avait jamais été réuni. Mais nous voudrions également connaître les intentions de l'État concernant le modèle économique et le financement des dépenses de fonctionnement de ce laboratoire. Il y va de l'avenir de cette université. Or, vous le savez, notre commission est également compétente en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Nous avons de nouveau échangé hier avec la présidente de l'université et nous souhaiterions maintenant connaître les garanties que l'État est prêt à lui apporter. Madame la ministre, le rôle du Sénat n'est jamais de ralentir l'examen d'un texte. Il s'agit toujours de veiller à en améliorer les dispositions. Dans le cadre d'une ordonnance, il nous revient d'obtenir les éclaircissements et les garanties nous permettant de nous assurer que l'habilitation législative sera convenablement utilisée. Notre vote de ce jour répondra, dans ces conditions, aux garanties que vous pourrez apporter à nos sujets de préoccupation. Je souhaite vivement qu'elles nous permettent de vous apporter dès aujourd'hui notre soutien à l'adoption de ce projet de loi. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues : « Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie. » En quelques mots, Aimé Jacquet a très bien résumé ce que représente le sport. C'est un vecteur de valeurs important dans une société. L'activité physique et la pratique sportive sont également cruciales en termes d'équilibre et de santé. La France compte des millions de licenciés sportifs s'inscrivant chaque année dans nos clubs. J'aime à dire que la vie associative est la plus belle école de la démocratie. Le sport représente des enjeux colossaux dans le monde, à la fois financiers ou encore d'influence. Bien souvent au cours de l'histoire, la politique et la diplomatie se sont invitées dans les rencontres sportives internationales dont la visibilité était importante. Le sportif doit être l'image d'un pays, d'une génération, le symbole d'une lutte et du courage. Le dopage dans le milieu sportif est un poison à large spectre, tant il véhicule des idées contraires à celles que je viens d'exprimer. La lutte contre le dopage est un combat de tous les instants. Les évolutions et les adaptations systématiques des législations nationales et internationales rendent efficace cette lutte. La révision du code mondial antidopage a cet objectif. Avant d'évoquer le projet de loi qui nous réunit cet après-midi, je souhaite associer à mes propos mon collègue sénateur du Nord, Dany Wattebled, qui a mis en valeur durant l'examen du dernier projet de loi de finances les impacts importants de la crise sur le milieu sportif et associatif dans notre pays. notre département du Nord, et plus largement dans la région des Hauts-de-France, nous sommes sensibilisés- cela vous surprendra peut-être -à la pratique sportive animale en compétitions et, donc, à la lutte contre le dopage animal. La pratique en compétitions nationales et internationales du sport colombophile est l'une des spécialités de notre territoire. La lutte contre le dopage lors de ces compétitions se fait dans le cadre de critères précis. Je sais que la lutte contre le dopage animal est aussi encadrée dans le code mondial antidopage et dans le code du sport français, et je m'en réjouis. Le projet de loi que nous étudions tend à habiliter le Gouvernement à mettre notre droit interne en conformité avec nos engagements internationaux en matière de lutte contre le dopage. Il me semble toutefois que le recours à une ordonnance est dommageable. Le sujet est délicat, et un débat parlementaire est toujours pertinent. Je comprends cependant les contraintes de temps dues à la situation actuelle et la nécessité d'adopter rapidement ce texte. Je salue l'exigence de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication dans ses demandes de précisions et de garanties. C'est indispensable. La France se prépare à accueillir des compétitions d'ampleur planétaire telles que la coupe du monde de rugby et les jeux Olympiques et Paralympiques. Chaque année, notre pays organise des rencontres de professionnels et d'amateurs. Le dopage n'y a pas sa place. Je salue la mise à jour par le code mondial antidopage des nouvelles catégories de substances interdites pour renforcer l'efficacité de la lutte, tout comme les modifications apportées concernant les sanctions, plus adaptables et flexibles. Selon moi, l'Agence française de lutte contre le dopage a une mission cruciale. Elle doit être suffisamment renforcée et les entraves doivent être levées. À cet égard, j'espère que les garanties demandées par la commission seront adoptées. très attaché à l'indépendance des organismes de contrôle, les moyens financiers des laboratoires, particulièrement dans la lutte contre le dopage, sont, à mes yeux, nécessaires. Il serait impensable que, par manque d'argent, le fonctionnement du nouveau laboratoire antidopage soit restreint ou simplement empêché. Il n'est pas envisageable de sous-traiter nos analyses et, donc, notre lutte à des organismes qui seraient moins chers sur le marché. Parce que le sport est une école de la vie, l'éducation joue le rôle de prévention. Les liens entre les échelons locaux, nationaux et internationaux sont précieux pour les règles antidopage et pour un sport propre, dont les valeurs restent celles de l'effort, du dépassement de soi, du courage et de l'esprit d'équipe. Tous les acteurs en présence doivent partager le même objectif contre le dopage. C'est une responsabilité commune. Sans la collaboration de tous, la lutte contre le dopage perd de son efficacité. Et sans la lutte contre le dopage, le sport perd son cap, celui de rassembler, d'émouvoir, de faire vibrer et de vivre ensemble. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte si les garanties demandées par le Sénat font l'objet de réponses concrètes.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France doit transcrire en droit interne la dernière version du code mondial antidopage, ce avant le 12 avril prochain. L'horloge tourne En cas de non-conformité, notre pays s'exposera à des sanctions, avec notamment l'interdiction de la participation de ses athlètes aux compétitions sportives internationales ou d'organisation d'épreuves sur son sol, ce que personne ne souhaite. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui tend donc à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, afin de répondre à l'urgence de la mise en conformité de notre droit national avec le nouveau code mondial antidopage. Pourquoi une telle urgence à agir maintenant, alors que le processus de révision du code mondial antidopage a été engagé en 2017 ?

Il nous faut donc légiférer maintenant, dans l'urgence, certes, mais aussi avec responsabilité. Sur le contenu de ce code antidopage, force est de le constater, il s'agit non pas d'une révolution, mais de quelques améliorations assez techniques et bienvenues visant à renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage. protection des personnes dénonçant des actes de dopage, protection bienvenue pour les lanceurs d'alerte ; la création d'une nouvelle catégorie de substances englobant les stupéfiants utilisés dans un contexte sportif ; et l'assouplissement des sanctions pour les sportifs de loisirs. Ces réformes, plutôt consensuelles, sont saluées par l'ensemble des acteurs. Toutefois, deux points en particulier ont retenu, en commission, l'attention du Sénat et l'ont empêché de voter le texte en l'état. Tout d'abord, concernant les pouvoirs confiés à l'Agence française de lutte contre le dopage, nous souhaitons que cette agence soit dotée de pouvoirs supplémentaires, notamment de convocation, d'audition et d'enquête. Ces pouvoirs d'enquête administrative sont d'ailleurs prévus par le nouveau code mondial antidopage. Ensuite, pour ce qui concerne le nouveau laboratoire antidopage, qui doit désormais être indépendant pour des raisons évidentes de lutte contre les conflits d'intérêts, des interrogations subsistent sur son modèle économique et les moyens nécessaires à son fonctionnement au sein de son organisme d'accueil, l'université

et du public qui nous regarde, concernant l'ordonnance que nous examinons aujourd'hui. Je le sais, vous avez mené un important travail de concertation avec l'AFLD, Paris-Saclay et nos rapporteurs. Le débat d'aujourd'hui est l'occasion d'en faire part publiquement. Mais ce projet de loi est aussi l'occasion d'aborder un sujet central, celui de la prévention. Madame la ministre, je crois comprendre que votre projet d'ordonnance prévoit simplement de confier aux fédérations sportives la tâche d'organiser des actions de prévention et d'éducation en lien avec votre ministère. L'intention est louable, mais elle reste encore déclarative. Le même reproche peut d'ailleurs être adressé au code mondial antidopage lui-même, qui fait de l'éducation et de la prévention des valeurs centrales, sans pour autant expliquer comment mettre celles-ci en oeuvre. On ne peut s'empêcher de voir dans la lutte contre le dopage les mêmes errements que ceux de nos sociétés dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Car les deux catégories de produits sont similaires, avec parfois les mêmes risques, les mêmes addictions et les mêmes dégâts pour la santé et l'intégrité physique. Ces questions ne seront pas simplement résolues en les limitant à la compétition du sport de haut niveau. Le dopage n'est pas un acte accompli uniquement par des athlètes soucieux de s'assurer les meilleurs classements. C'est une pratique présente partout dans le sport, depuis les amateurs qui se procurent des produits douteux sur internet jusqu'aux sportifs de haut niveau aidés par des équipes médicales peu scrupuleuses. Tous les sports, tous les milieux, sont concernés. Ainsi, comme souvent, le tout-répressif montre-t-il ses limites. Il nous faut de l'éducation, de la prévention, mais aussi de l'accompagnement sanitaire, et des politiques de sortie de l'addiction.

Loin d'être superflu, le code mondial antidopage est l'outil qui permet d'harmoniser les politiques, les règles et les règlements antidopage des organisations sportives et des autorités publiques internationales. Assorti de huit standards, ce code est un outil nécessaire pour protéger le sport et son éthique des différentes formes de dopage. Il est aussi, me semble-t-il, un exemple rare de coopération politique efficace à l'échelle mondiale. Le Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique, les fédérations internationales, les organisations nationales et régionales antidopage : autant de signataires d'un code mondial antidopage qui fait consensus, puisque près de 700 organisations sportives l'ont accepté. Mais vous n'êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que ce code, comme tant d'autres, n'a jamais été conçu pour être un outil statique. Au contraire, il doit évoluer. Après deux révisions, en 2007 puis en 2013, le processus de révision pour 2021 est arrivé à son terme avec l'adoption à l'unanimité du code révisé en novembre 2019. Cela ne vous aura pas échappé le code 2021 est donc entré en vigueur le 1 janvier 2021. Pourtant, si les instances françaises sont bien évidemment signataires du code, sa mise en oeuvre est aujourd'hui bloquée. La raison en est simple : les règles issues de la nouvelle version du code n'ont pas été transposées en droit interne. Autrement dit, depuis le 1 janvier, le droit français n'est plus en conformité avec la nouvelle version du code

agir rapidement ! Sans plus attendre, nous devons autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Mes chers collègues, il me semble qu'une telle autorisation est nécessaire, pour deux raisons. Elle est nécessaire parce que nous devons permettre au Gouvernement d'assurer la mise en conformité du droit interne avec les nouvelles règles dans les plus brefs délais. N'aurions-nous pas honte d'être l'objet d'une sanction alors que notre pays s'apprête à organiser, entre autres, la coupe du monde de rugby en 2023 et les jeux Olympiques en 2024 ? Cela n'est pas sérieux, et nous méritons mieux. ni l'héritage de notre histoire sportive ni les retrouvailles tant espérées entre le sport et les Français. Elle est nécessaire, également, parce que notre pays doit poursuivre intelligemment sa lutte contre le dopage. Grâce aux avancées majeures proposées dans le code mondial antidopage peut dès maintenant mettre à jour son action en modulant davantage les sanctions et en améliorant la protection des lanceurs d'alerte. La France doit entamer une mise à jour à la fois formelle et intellectuelle. Jusqu'à présent, la stratégie adoptée n'était pas optimale. Ces dernières années, la réglementation avait eu pour effet de dessaisir les fédérations de lutte antidopage. Le projet de loi que nous votons cet après-midi permet de créer une politique de lutte contre le dopage axée sur la collaboration entre les différents acteurs du monde du sport : une lutte transformée, avec le collectif Comment ? En définissant un nouveau statut pour le laboratoire d'analyses antidopage, qui sera dorénavant un organe distinct de l'Agence française de lutte contre le dopage. L'objectif est de garantir l'indépendance administrative et opérationnelle des laboratoires vis-à-vis des agences antidopage. Dans cette lutte, il n'y a pas de place pour les conflits d'intérêts. Le laboratoire de Châtenay-Malabry, qui est depuis 2006 un département de l'Agence française de lutte contre le dopage, ne peut plus être administré par celle-ci. Mme la ministre l'a rappelé : le projet d'intégration du laboratoire au sein de l'université Paris-Saclay est en très bonne voie, puisque le transfert prendra effet le 1 janvier 2022. Le projet de loi autorise en outre le Gouvernement à renforcer les pouvoirs de l'Agence française de lutte contre le dopage. Avec des prérogatives élargies et un dispositif de recueil d'informations simplifié, l'AFLD sera mieux armée pour combattre les comportements dopants, protéger davantage les sportifs contre les tentations offertes en ligne et réprimer plus efficacement les violations. les délais impartis et la situation dans laquelle nous sommes, le groupe RDPI appelle à la responsabilité. Le Gouvernement a apporté les garanties demandées par la commission par la voix de Mme la rapporteure voter contre ce projet de loi retarderait l'échéance d'une mise en conformité déjà lambine. Pire encore, cela rendrait légitime la concrétisation du risque de sanctions à venir. le sujet de l'éthique sportive doit l'emporter sur toute autre considération politique. C'est pourquoi nous voterons pour ce projet de loi et vous appelons à faire de même. La

avec la lutte contre le dopage et la conformité au code mondial antidopage, nous sommes loin du sport-santé et de l'exercice physique recommandé pour tous. Le sport est un puissant promoteur de l'exercice physique pour tous. Les disciplines sportives ajoutent à cela une dimension pédagogique la codification de leurs règles du jeu. L'apprentissage et les entraînements développent le goût de l'effort, le dépassement de soi, dans le respect des règles, des adversaires, des arbitres et des partenaires. La communion avec les spectateurs renforce la fraternité, et la dimension esthétique de certaines pratiques sportives embellit la vie. Mais si une alimentation saine, une réhydratation, des compléments vitaminiques sont recommandés, les limites d'une bonne hygiène de vie ne doivent pas être franchies par la tentation de créer un « humain augmenté » par le dopage. Les limites doivent être claires et reconnues. Les franchir est une tricherie et un très mauvais exemple pour une jeunesse dont le sport participe à l'épanouissement. Le code mondial antidopage est conçu pour ça, et il est important de mettre notre droit interne en conformité avec ses règles, au titre de l'adhésion de la France à la convention internationale contre le dopage dans le sport. Cette convention donne une force contraignante aux décisions et aux règles édictées par l'Agence mondiale antidopage. La financiarisation de la société et la commercialisation du sport poussent à bien des abus et à bien des fautes. Il convient donc de donner des moyens efficaces d'enquête à l'Agence française de lutte contre le dopage. L'évolution des techniques de dopage, l'utilisation de nouvelles substances imposent de faire évoluer les règles et les moyens de contrôle.

C'est pourquoi, avec la commission, nous attendons des réponses concrètes sur le pouvoir d'enquête administrative de l'AFLD, signataire du code mondial antidopage,

cependant d'une décision récente des États-Unis, le, adopté en novembre dernier, qui assoit l'extraterritorialité du droit américain. Les autorités américaines peuvent désormais poursuivre toute personne impliquée dans un système international de dopage, quelle que soit sa nationalité. Comment la France se positionne-t-elle face à une décision qui pourrait saper la capacité de l'Agence mondiale antidopage à accomplir sa mission de régulateur global ?

Plus vite, plus haut, plus fort », cette maxime qui fonde l'esprit olympique et sportif est un appel au dépassement de soi. Malheureusement, elle semble avoir été mal comprise par certaines et certains. Premièrement, s'il est bien évidemment question d'éthique, il est aussi question de santé publique. On ne compte malheureusement plus, depuis le cycliste Arthur Linton en 1896, les morts consécutives à l'absorption de produits dopants. Deuxièmement, loin de réduire les personnes dopées à de « mauvais joueurs », il faut aller aux sources du dopage. C'est d'autant plus essentiel qu'il n'est plus question d'une pratique propre au haut niveau : le dopage se retrouve à tous les étages du mouvement sportif. En ce sens, le devoir de prévention vaut lui aussi à tous les niveaux. La professionnalisation du sport a entraîné

tous ces éléments participent indirectement à la peur de la mauvaise performance et peuvent, malheureusement, être un terreau favorable à la triche. Troisièmement, on constate que les enjeux du sport dépassent largement aujourd'hui la question du divertissement, et même de l'économie. Ne faut-il pas voir dans les systèmes institutionnalisés de dopage

Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est le bienvenu. Je sais, madame la ministre, que vous auriez souhaité qu'il soit adopté plus tôt ; nous aussi, évidemment. Je sais aussi, et je vous en sais gré, que vous avez souhaité un dialogue constant avec la représentation nationale afin de faciliter son adoption. Toutefois, il souffre encore de certaines limites, à propos desquelles votre engagement reste uniquement oral. tout d'abord les pouvoirs de l'AFLD, malgré les garanties que vous avez apportées à l'Agence depuis notre réunion de commission, l'ordonnance reste extrêmement floue. Pourtant, les demandes de l'AFLD sont plutôt simples : elle souhaite être dotée des prérogatives qui lui permettraient d'exercer les missions pour lesquelles elle a été créée en 2006.

D'une part, la quasi-totalité des manquements aux règles antidopage ne sont pas repérables par analyse. D'autre part, il importe, si l'on veut faire de l'AFLD le phare français de la lutte contre le dopage, de lui donner les moyens de mener ses enquêtes dès qu'un faisceau d'indices se présente.

Quand pouvons-nous espérer que soit créé un service commercial lui permettant de facturer ses prestations ? Son chiffre d'affaires sera-t-il suffisant pour maintenir et même amplifier son activité ? Si non, qui viendra le soutenir ? Vous le voyez, nous avons encore beaucoup de questions. Et selon les réponses qui y seront données, c'est toute la réussite du projet qui sera ou

à Katowice, et un an après le dépôt de ce projet de loi, nous soyons encore un peu dans le flou. Le dialogue mené ces quinze derniers jours semble avoir été plus intense et plus productif qu'au cours des douze mois précédents. Malgré ses limites, le groupe communiste pour deux raisons. Premièrement, parce que l'urgence nous l'impose : nous n'avons d'autre choix que de faire avec l'intransigeance bienvenue de l'AMA. Deuxièmement, parce que ce texte contient aussi de vraies avancées, en matière d'individualisation et de proportionnalité des sanctions ou encore de protection des lanceurs d'alerte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis l'adoption du premier code mondial antidopage, en 2003, deux versions l'ont fait évoluer, en 2009 et en 2015.

Rappelons que ce texte d'origine privée, donc sans effet direct, doit néanmoins être appliqué par la France, dans la mesure où nous sommes liés par la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l'Unesco du 19 octobre 2005, qui prévoit notamment, dans son article 3, que les États parties s'engagent à « adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le code [mondial antidopage] Le but du code est de promouvoir la lutte antidopage par l'harmonisation universelle des principaux éléments de cette lutte. L'objectif est de protéger le droit fondamental des sportifs à participer à des activités sportives sans dopage, de promouvoir la santé et de garantir aux sportifs du monde entier l'équité et l'égalité dans le sport. est aujourd'hui en retard ; nous pouvons dire que nous nous trouvons dans le trio de queue européen en ce qui concerne la transposition en droit interne des prescriptions du code mondial antidopage.

Je sais néanmoins l'attachement de la France à respecter ses engagements internationaux et, plus largement, à figurer parmi les nations actives pour la préservation de l'intégrité sportive et la protection des sportifs. À ce titre, la France, sur le fondement, notamment, du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avait engagé un vaste plan de modernisation de son dispositif de lutte contre le dopage visant à mieux prévenir ce fléau mais aussi à harmoniser son organisation avec les standards de l'Agence mondiale antidopage. Elle avait ainsi modifié par ordonnance la procédure disciplinaire en vigueur en matière de lutte antidopage. Or, malheureusement et encore une fois dans l'urgence, nous sommes sommés de nous mettre en conformité avec les normes édictées par l'AMA avant le 12 avril, ce qui est demain Cette transposition permettra de mettre en conformité le droit interne avec les principes du code mondial antidopage et ainsi d'intégrer les toutes dernières évolutions concernant la création de nouvelles violations des règles antidopage, la possibilité de moduler davantage les sanctions ou encore l'amélioration de la protection des lanceurs d'alerte. L'un des enjeux majeurs est aussi d'assurer la séparation organique du laboratoire d'analyses antidopage d'avec l'AFLD, dans la continuité du processus de modernisation lancé avec la construction d'un nouveau laboratoire. Enfin, cette transposition permettra de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le dopage, en facilitant le recueil d'informations par l'AFLD et la coopération entre les acteurs de cette lutte. On attend donc de notre chambre haute qu'elle vote conforme ce texte pour répondre à cette nécessité de célérité- et je tiens à saluer l'excellent travail de notre rapporteure, Elsa Schalck. Notre attente était forte à l'égard des engagements de l'État, qui se devaient d'être pragmatiques compte tenu des besoins inhérents à cet important chantier. Le dopage est un véritable fléau qui gangrène le sport, professionnel et amateur, et les moyens d'y faire face doivent être à la hauteur de la tâche.

et, d'autre part, sur la structure même des pouvoirs d'enquête administrative accordés à l'AFLD- je citerai notamment le pouvoir de convocation et la faculté d'utiliser une identité d'emprunt par internet, pouvoirs dont disposent, je le rappelle, d'autres autorités indépendantes comme l'Autorité des marchés financiers. En effet, aujourd'hui, la capacité d'action de l'AFLD se limite à un pouvoir de contrôle la réalisation de prélèvements biologiques

les comportements répréhensibles, dans un but de protection des sportifs avant tout. Nous attendons maintenant que vous confirmiez devant la représentation nationale les engagements du Gouvernement lors de l'examen des amendements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'harmonisation internationale des régimes de contrôle et de sanction du dopage est fondamentale. Le système ne peut être accepté et respecté par la totalité des acteurs du monde sportif que si chacun est soumis aux mêmes règles, tant dans le cadre des épreuves nationales que dans À quoi servirait l'application d'un plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes dans les activités physiques et sportives, et à quoi servirait notre politique de contrôle et de sanction, si à la moindre compétition internationale nos athlètes se trouvaient confrontés à des adversaires enfreignant la loi et violant le principe de l'équité dans la compétition ? Le talent et le travail doivent demeurer les moteurs de la performance. Le présent projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance aux modifications législatives nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage, l'échelon international fixant le cadre de la réflexion et de la coopération entre les différentes agences étatiques antidopage. La France, qui figure parmi les pays leaders dans la lutte contre le dopage, a toujours veillé à créer les conditions juridiques nécessaires à la mise en oeuvre complète du code mondial antidopage, édicté depuis 2003 par l'Agence mondiale antidopage et qui fait régulièrement l'objet d'évolutions. constitue la base juridique s'imposant à l'ensemble des pays signataires de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée en 2005 sous l'égide de l'Unesco. La création de l'AMA et la rédaction du code mondial antidopage ont marqué une étape historique dans l'histoire des compétitions.

dernière est portée par l'AMA, dont les décisions sont parfois critiquées mais dont le rôle est incontournable. L'AMA doit être défendue et consolidée toujours davantage, notamment financièrement. Elle est financée à parts égales par le CIO, d'une part, et les gouvernements, Mais alors que 191 États ont adopté en 2005, à l'unanimité, la convention internationale de l'Unesco contre le dopage dans le sport, le budget de l'AMA s'élève seulement à 32 millions d'euros, soit 5 % du seul budget du PSG La loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs avait par avance mis la législation en adéquation avec la première version du code mondial antidopage. Puis trois révisions dudit code entraînèrent des mises en conformité de sa partie législative, successivement intervenues par voie d'ordonnance en 2010, 2015 et 2018. Dans la continuité de cette mise en conformité régulière, il nous revient aujourd'hui d'adapter le droit national à la version du code mondial adoptée lors de la conférence mondiale de Katowice de 2019, version entrée en vigueur depuis le 1 janvier 2021. La réforme organisationnelle se poursuit donc, étape après étape. Mais le retard pris par la France a conduit l'AMA à lui adresser un rapport de mesures correctives qualifiant de « critique » cette irrégularité et lui accordant un délai de trois mois, soit jusqu'au 12 avril prochain. Il expose le pays à des sanctions lourdes de conséquences ; la France doit respecter ses engagements internationaux. Mettons-nous un instant à la place du sportif de haut niveau et de son encadrement ; ils sont soumis à de multiples contraintes : contrôles réguliers, inopinés ou en compétition, localisation par le système dit « Adams » Ils ne comprendraient pas que les efforts consentis soient contrariés par des difficultés, voire des entraves, à caractère administratif et institutionnel. D'où notre niveau d'exigence élevé quant à l'accomplissement des missions de l'AFLD, aux moyens qui lui sont accordés et à l'application du code mondial. La mise en oeuvre de telles sanctions aurait également des répercussions négatives en termes d'image dans la perspective de l'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 et des jeux Olympiques de 2024. L'enjeu est donc majeur pour la France, qui, précisément, s'est fixé des objectifs pour 2024, en nombre de médailles ou en augmentation du nombre de pratiquants ; elle doit également se fixer de hautes ambitions sur les plans déontologique et éducatif. Concrètement, les nouveaux standards internationaux déclinés dans l'unique article de ce projet de loi offrent de réelles avancées. Au sein de la commission d'enquête parlementaire sur l'efficacité de la lutte contre le dopage, nous avions identifié les obstacles auxquels cette lutte était confrontée : la loi du silence, l'internationalisation des trafics, quarante-huit heures, on peut se faire livrer de l'érythropoïétine (EPO) à domicile -et, parfois, les pressions politiques et les complicités institutionnelles, mais aussi les difficultés de détection de certains produits, l'apparition de nouveaux protocoles très individualisés, un paysage audiovisuel peu motivé par des campagnes de prévention, un manque d'informations transmises aux sportifs de haut niveau. Ces difficultés demeurent, mais le contour des ordonnances envisagées dans ce projet de loi d'habilitation représente des avancées dans divers domaines : l'éducation et la prévention, la coordination des acteurs, la prise en compte des preuves non analytiques, l'individualisation des sanctions, l'actualisation de la liste des produits concernés, l'autonomisation des laboratoires, la protection des individus qui dénoncent des faits de dopage aux autorités, c'est-à-dire des lanceurs d'alerte ; tout cela va dans le bon sens. Mais deux évolutions ont particulièrement alerté notre commission, au point que celle-ci a rejeté le texte lors de son examen le 3 février dernier,

revient à acter sa séparation d'avec l'AFLD, qui, depuis 2006, l'administrait. Alors que le laboratoire et ses personnels doivent rejoindre la faculté de pharmacie de l'université Paris-Saclay au 1 novembre prochain, cette intégration semble souffrir d'un manque d'ingénierie et de moyens déployés. Le laboratoire assumera lui-même le coût de son fonctionnement à partir de la rémunération des prestations qu'on lui achètera, de recettes extérieures, mais également de la subvention d'équilibre du ministère des sports, qui lui permettront de financer ses investissements. Il convient donc, madame la ministre, d'apporter les éclaircissements et les garanties indispensables à la réussite de ce projet. J'ajoute que les opérations de recherche et développement, éléments structurants de la lutte antidopage, apparaissent peu dans ce texte de mise en conformité. Le second point d'achoppement concerne l'impossibilité pour l'AFLD, au regard du droit français actuel,

le Parlement a légiféré à de nombreuses reprises, avec une continuité évidente dans la recherche de l'efficacité. Cette action s'inscrit dans la durée, la France devant continuer à jouer un rôle moteur dans cette lutte, traduction d'une vision humaniste du sport. Je rappelle que la généralisation du passeport biologique et du suivi longitudinal est due à un amendement sénatorial. Plus globalement, la lutte antidopage progresse, mais tout relâchement serait coupable. S'il semble de plus en plus difficile de passer entre les mailles du filet, les substances et les protocoles indécelables menacent toujours. Nous sommes dans un système de tolérance zéro où la finalité est claire : l'éradication des substances prohibées. aussi reconnaître que la suspicion de dopage peut parfois ternir l'image d'une discipline sans preuve objectivement démontrée. La relation sport-dopage est rythmée de drames, d'affaires, de scandales, depuis les jeux Olympiques antiques. Pour la période contemporaine, le décès du cycliste Tom Simpson, les affaires Festina, Puerto, Pistorius, Ferrari, Balco, le scandale Armstrong, le dopage d'État aux jeux Olympiques de Sotchi, les démêlés judiciaires de la Juventus de Turin, pour ne citer qu'eux, furent autant de révélateurs fracassants d'une réalité encore souvent dominée par le secret et le refus d'assumer ses responsabilités. Les sportifs tricheurs ont souvent bénéficié d'un manque de transparence et de coopération entre les parties concernées, menaçant parfois la crédibilité même de la lutte antidopage. La valorisation du rôle des sportifs repentis, véritables briseurs d'omerta, va dans le sens d'une meilleure connaissance du phénomène du dopage. Les valeurs du sport, toujours prônées, mais souvent perverties, comptent la loyauté dans leur arsenal, mais également la sécurité sanitaire du pratiquant. Le dopage est bien un enjeu de santé publique. Il n'est pas lié à tel ou tel sport puisqu'il concerne l'homme face à la compétition. Mais les mentalités évoluent : sont de moins en moins nombreuses les personnes qui pensent que le dopage n'existe pas ou n'est pas un problème dans le sport, ou qui remettent en cause la nécessité, voire les principes, de la lutte antidopage, ou bien encore qui veulent garder les yeux fermés sur ces pratiques délictuelles pervertissant la loyauté des compétitions. Le sujet n'est plus vraiment tabou. Le combat contre le dopage est un combat juste ; nous devons en tirer les conséquences en donnant des moyens financiers et juridiques à l'ensemble des acteurs impliqués- et ils sont nombreux. Madame la ministre, sur les trois sujets qui méritaient à nos yeux un éclaircissement et des garanties, nous prenons acte des avancées enregistrées ces derniers jours. Nous sommes prêts à voter ce texte.

Je tiens ici à témoigner de la qualité des auditions et de votre volonté de partager avec l'ensemble de vos collègues les problématiques soulevées lors de ces échanges. Je souhaite aussi remercier le président de notre commission, qui s'est fortement mobilisé sur ce dossier. C'est grâce à ce travail précis et empreint d'une volonté de coconstruction que nous abordons ce débat. Ce projet de loi, qui était présenté comme une simple formalité pour assurer la conformité de notre code antidopage aux principes du code mondial antidopage, a fait apparaître quelques points qui méritent des réponses et des engagements précis du Gouvernement. Nous sommes bien conscients que ce texte est d'une absolue nécessité ; nous le devons à nos athlètes et para-athlètes, qui portent chaque jour les couleurs de la France au plus haut niveau international. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce qu'ils ne puissent plus participer aux différentes compétitions en raison d'un manquement de la France. De De nouvelles dispositions vont permettre plusieurs avancées en termes d'antidopage, notamment en renforçant la coopération entre les acteurs. Ce point me paraît central et attendu, car il permettra d'accroître la responsabilisation de tous les acteurs, notamment des fédérations. celles-ci souhaitent s'impliquer plus largement dans la lutte contre le dopage, il convient de leur en donner les moyens nécessaires. La lutte antidopage est un combat commun de chaque instant, et nous devons être intransigeants sur ce sujet.

il nous a été indiqué à plusieurs reprises que nous étions dans l'obligation de voter conforme ce projet de loi, parce qu'il y a urgence à agir, que l'Agence mondiale antidopage (AMA) a laissé à l'AFLD un délai de trois mois pour se mettre en conformité, que la France fait partie des trois derniers pays à ne pas être en règle, qu'en cas de manquement le sport français serait sanctionné avec un risque d'exclusion de nos athlètes des compétitions internationales. Alors que nous allons organiser la coupe du monde de rugby en 2023 et les jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, cela ferait tache ! Le Gouvernement a laissé traîner le sujet, ce qui est regrettable. Car, avec les délais qui nous sont aujourd'hui imposés, c'est une nouvelle fois une occasion manquée d'avoir un véritable débat de qualité sur la lutte contre le dopage dans notre pays, sur les moyens qui y sont affectés et sur notre ambition commune en la matière. Ensuite, sur le fond. Lors des différentes auditions, nous n'avons pu que constater que de nombreux points restaient à régler en matière d'antidopage : sur les moyens, le financement, les partenariats, l'organisation, la collaboration entre les différentes instances, etc. Nous le constatons donc, la situation est aujourd'hui est plus compliquée qu'il n'y paraît. Je ne vais pas reprendre tous les aspects extrêmement bien évoqués par notre rapporteure et que je partage pleinement. Mais je voudrais revenir sur deux points déjà relevés par mes collègues et sur lesquels- vous les avez déjà abordés

Par ailleurs, nous avons besoin de garanties concernant le nouveau laboratoire antidopage. L'ordonnance doit définir le nouveau statut du laboratoire, dont le code mondial antidopage prévoit qu'il doit être dorénavant séparé de l'Agence. Ce sera chose faite avec le nouveau laboratoire intégré au sein de l'université Paris-Saclay. Cette évolution est tout à fait essentielle pour s'assurer de son entière indépendance, administrative comme opérationnelle. Des engagements doivent être pris à l'égard de l'université non seulement sur la compensation des charges, en particulier s'agissant des fonctions support, mais aussi sur le régime de responsabilité applicable au laboratoire, puisque celui-ci devrait être rattaché à la faculté de pharmacie tout en conservant son autonomie. Ensuite, il faut apporter des garanties quant à la pérennité de ces financements. Nous voulions pour cela être assurés que, au-delà du transfert par l'AFLD des moyens existants du laboratoire à l'université, votre ministère sera vigilant à définir dans les prochains mois le futur modèle de financement du laboratoire et sa programmation pluriannuelle, ce qui inclut en particulier l'équipement en matériel technique de pointe surtout dans la perspective des jeux de 2024. Vos propos au début de la discussion générale nous ont rassurés, au moins sur ces points. J'ai déposé un amendement pour prévoir que le modèle économique et les moyens nécessaires au fonctionnement du nouveau laboratoire seront déterminés dans le cadre d'une convention signée entre l'État et et l'organisme d'accueil, en l'espèce l'université Paris-Saclay. La clarification de ce modèle économique est un point essentiel auquel nous tenons ; là encore, j'espère que vous pourrez, madame la ministre, vous engager fermement sur ce point. Je tiens toutefois à nous féliciter, car nos doutes ont d'ores et déjà produit une partie des effets escomptés avec la convocation du comité de pilotage, qui ne s'était encore jamais Vous l'aurez compris, notre démarche collective correspond à la volonté affichée du Sénat d'être constructif. Nous prendrons nos responsabilités, mais nous soulignons également celles qui incombent au Gouvernement. J'espère cependant que nos débats permettront d'avancer sur le sujet, et que nous aurons l'occasion de rassurer les acteurs de la lutte antidopage de notre pays.

à l'AFLD pour lui permettre d'exercer ses nouvelles missions prévues par le code mondial antidopage, parmi lesquelles figurent, en particulier, un pouvoir de convocation et d'audition et la capacité à utiliser une identité d'emprunt sur les sites internet. Madame la ministre, je vous remercie de nous confirmer les engagements du Gouvernement que vous avez évoqués lors de la discussion générale.

une relation différente entre l'État et les fédérations sportives. Le contrat de délégation « nouvelle génération » permettra aux fédérations de s'engager concrètement dans un plan d'action, avec des indicateurs, notamment pour suivre le plan de lutte contre le dopage : nous aurons à nos côtés des acteurs engagés.

à la pointe de la technologie, afin de permettre un travail dans les meilleures conditions possible, pour que la France redevienne le leader mondial en matière de lutte contre le dopage, ce qui était le cas il y a encore quelques années.

acté un échéancier, avec un comité de pilotage qui se réunira régulièrement et sera accompagné par l'inspection générale. Nous pouvons d'ores et déjà vous assurer que nous irons dans le sens que vous évoquez, c'est-à-dire une budgétisation pluriannuelle et un soutien aussi bien aux fonctions support qu'aux investissements, pour que ce laboratoire collabore en intelligence et en pertinence avec la faculté de pharmacie à laquelle il sera désormais rattaché.

La séance est reprise. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement. Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 29 de notre règlement. Nous avons observé, depuis un certain temps, des recours multiples et variés à des cabinets d'avocats pour rédiger la loi

notre Parlement. C'est la raison pour laquelle je souhaitais faire ce rappel au règlement de façon que nous puissions avoir au sein de notre Haute Assemblée un débat sur cette question. En effet, il me semble que, au fur et à mesure que le Gouvernement confie ces fonctions à des cabinets extérieurs, nous perdons

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd'hui un projet de loi qui ratifie quatre ordonnances, toutes prises en application de la loi du

Nous nous rappelons tous, et vous particulièrement dans cet hémicycle, du contexte difficile dans lequel nous avons dû légiférer en mars dernier. Quand le Gouvernement avait demandé au Parlement d'être habilité à prendre ces ordonnances, nous étions face à un scénario inouï : un virus inconnu avait mis notre pays, et même notre planète, à l'arrêt. Je me souviens, alors que j'étais députée lors de la présentation de ces ordonnances au Parlement, de l'agilité à toute épreuve de notre administration pour faire face à cette urgence inédite. Grâce à elle, nous avons pu, en quelques jours, mettre en place un des systèmes les plus protecteurs du monde pour nos entreprises et pour l'emploi. En quelques jours, notre système était prêt à faire face de façon efficace : près d'un an plus tard, notre protection économique tient encore, grâce à son adaptation constante notamment permise par les travaux des parlementaires. Il est des anniversaires plus heureux que d'autres. Je veux néanmoins saluer et remercier tous ceux qui, au sein de notre administration, ici et en services déconcentrés, ont accompagné au quotidien les parties prenantes de notre économie. Vous le savez, n'est pas encore révolu, et les mesures contenues dans ces ordonnances ont un rang législatif. Il convient donc que le Parlement s'en saisisse et les ratifie. Après l'adoption de ce projet de loi de ratification,

qui ont bénéficié de près de 12 milliards d'euros en 2020. Ce soutien est inégalé. Il a permis à nos entreprises de garder la tête hors de l'eau et le permet encore aujourd'hui, après plusieurs élargissements importants décidés au fil des mois. Il vous est également proposé de ratifier une autre de nos réponses aux importants besoins de trésorerie des entreprises, à savoir l'ordonnance relative à l'octroi d'avances en compte courant par les organismes de placement collectif de capital investissement. Le but était de permettre aux acteurs du capital investissement de renforcer leur soutien aux entreprises de leur portefeuille, en complément des importants moyens publics mobilisés. avec cette ordonnance, les fonds de capital investissement ont pu dépasser temporairement le plafond légal qui restreint, en temps normal, leur capacité à consentir des avances en compte courant aux entreprises dont ils sont actionnaires. La ratification de cette ordonnance permettra de confirmer le délai dont bénéficient les acteurs pour revenir au régime de droit commun, d'ici au 30 juin 2022. La même logique de régime dérogatoire permettant de renforcer le soutien aux entreprises prévaut pour la ratification de l'ordonnance du 17 juin 2020 relative à la commande publique. Cette dernière introduit, au sein du droit de la commande publique, des outils permettant de soutenir les opérateurs économiques les plus fragilisés par la crise.

à l'apurement de leur passif avec la conclusion de nouveaux contrats. Aussi, elle ouvre aux PME un accès privilégié aux marchés publics globaux, en fixant à 10 % la part d'exécution minimale qui sera confiée

de proximité. Nous sommes convaincus que la relance passera par ces entreprises de nos territoires et que la commande publique peut, et surtout doit, être un accélérateur de la relance. C'est la raison pour laquelle, jusqu'au 31 décembre 2023, la capacité économique et financière des candidats aux marchés publics ne pourra être évaluée sur les périodes où ils auraient pu directement subir les effets de la crise sanitaire. Les dérèglements économiques de la période sont le fait du virus, pas du chef d'entreprise- il est toujours bien de le rappeler. Enfin, je voudrais m'arrêter un moment sur l'article 3 du présent texte de loi, qui ratifie l'ordonnance portant réorganisation de notre banque publique d'investissement, Bpifrance. Pour rappel, l'opération de réorganisation du groupe Bpifrance consiste à ce que l'ancienne filiale bancaire, Bpifrance Financement SA, absorbe la société faîtière Bpifrance SA, et devienne dès lors la nouvelle société mère du groupe. Cette opération a notamment pour but de donner à l'établissement de crédit une solvabilité supplémentaire, laquelle lui permettra de jouer pleinement son rôle-

de renforcer la sécurité juridique des dispositifs qui viennent en aide à nos entreprises, dans un contexte économique particulièrement difficile depuis bientôt un an, et surtout de permettre à celles-ci d'aborder la reprise et la relance de la meilleure façon possible. je vous remercie

le projet de loi qui nous est soumis a pour objet de ratifier plusieurs ordonnances prises par le Gouvernement, dans le cadre de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie concernent le fonds de solidarité, des adaptations du droit applicable à la commande publique, les avances en compte courant des fonds d'investissement et, surtout, la réorganisation de Bpifrance

Je veux saisir cette occasion pour rappeler que le soutien apporté par le fonds de solidarité aux petites et moyennes entreprises a été tout à fait vital. Les derniers chiffres sont là pour le démontrer : plus de 15 milliards d'euros ont ainsi été accordés à près de 2 millions d'entreprises. En complément du fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État (PGE), l'activité partielle et les exonérations de cotisations sociales constituent des leviers déterminants pour sauver l'économie et l'emploi ; je souhaite y revenir

Enfin, les secteurs les plus touchés par les restrictions ont bénéficié d'une exonération de charges patronales. Le coût de ce dispositif, lui aussi nécessaire, s'élève à 4 milliards d'euros pour 2020. Je tiens à le rappeler, l'ensemble de ces mesures étaient absolument nécessaires et ont démontré leur efficacité. évidemment, des interrogations demeurent : dans un contexte de pandémie qui perdure, les entreprises seront-elles en mesure de rembourser la dette covid qu'elles auront accumulée pour traverser la crise sans affecter leur capacité de rebond ?

temporaires -en matière de commande publique. Trois évolutions principales sont envisagées : permettre aux entreprises faisant l'objet d'un plan de redressement judiciaire de se porter candidates aux marchés publics et aux contrats de concessions étendre à l'ensemble des contrats globaux du code de la commande publique le critère d'une part minimale de 10 % d'exécution du contrat réservée aux PME, ce qui est très important ; et imposer aux acheteurs publics de ne pas tenir compte de la baisse de chiffre d'affaires liée à la crise des candidats aux marchés publics ou contrats de concession. Ces mesures sont utiles ; elles doivent permettre aux acheteurs publics, en particulier aux collectivités locales, de soutenir les entreprises et l'emploi dans tous les territoires. Si les mesures de l'article 4 sont de nature plus technique, la logique est la même : il s'agit d'activer des leviers juridiques pour venir en aide aux entreprises. Ainsi, il est proposé de ratifier l'ordonnance du 17 juin

La première est d'ordre purement juridique : l'ampleur de l'ordonnance est plus large que le champ de l'habilitation accordée en mars dernier. La seconde est d'ordre plus opérationnel, la sécurisation législative de l'ordonnance étant de nature à rassurer tant les investisseurs que la Banque centrale européenne.

de Bpifrance Participations et de multiplier ainsi par plus de cinq le montant de ses fonds propres, renforçant considérablement ses capacités de financement de l'économie ; d'autre part, elle simplifie l'organisation et la gouvernance de la structure. C'est pourquoi, mes chers collègues, cette réorganisation, qui permet de renforcer le soutien de l'économie dans un moment où ce soutien est absolument nécessaire, bénéficie de l'appui de notre commission. Toutefois, les modalités retenues par le Gouvernement emportent plusieurs conséquences, sur lesquelles je souhaite revenir. La première concerne la détention du capital.

et à 9 % par des investisseurs privés, essentiellement des banques françaises. L'absorption par Bpifrance Financement de la société de tête se traduit donc par une modification des conditions de détention 98,6 % du capital est détenu à parité par l'État et la Caisse des dépôts, et 1,4 % par des investisseurs privés. L'ordonnance, qui date de juin dernier, fixait un plancher de 95 % à la détention publique. Ce taux, retenu en amont de l'opération, a permis de préserver une certaine souplesse, alors que les valorisations respectives des deux entités fusionnées n'étaient pas encore définitivement arrêtées.

L'entité de tête pourra ainsi s'endetter sans que cela soit comptabilisé dans les indicateurs maastrichtiens. Bpifrance continuera donc de bénéficier de conditions favorables grâce à la garantie de l'État et pourra ainsi augmenter la dotation de Bpifrance Participations sans conséquence sur le solde public. Je tenais à souligner cette donnée importante. Enfin, un dernier point point a retenu mon attention ; les fonds de garantie dédiés aux prêts aux PME sont abondés, depuis plusieurs années, par des redéploiements de crédits et des recyclages de dividendes. de dividendes. La nouvelle organisation issue de la fusion pourrait conduire à accroître ces pratiques, qui peuvent sembler en contradiction avec le principe d'universalité budgétaire, lequel veut que le Parlement ait à se prononcer sur l'usage des deniers publics.

Les marges de manoeuvre qui avaient été données au Gouvernement en début de crise sanitaire, face à l'urgence de la situation, ne doivent pas empêcher le contrôle démocratique de la représentation nationale ni faire glisser le régime sanitaire qui nous est imposé depuis désormais un an vers un régime d'ordonnances. Non seulement l'état d'urgence doit faire l'objet de ce contrôle parlementaire,

de rappeler que la concertation et le débat démocratique ne sont pas exclusifs d'une décision tout à la fois efficace et proportionnée, sauf à remettre en cause les piliers mêmes de notre République.

Néanmoins, permettez-nous de le souligner, les conditions pour bénéficier de ce fonds, certes élargies à l'automne dernier, ont fait perdre de la clarté et de la visibilité à ce dispositif, dont l'impact pourrait être beaucoup plus important si vous acceptiez sa territorialisation ; cela cela permettrait un fonctionnement plus souple et la prise en charge de situations non prévues dans le cadre législatif et réglementaire actuel, et cela permettrait d'accompagner plus équitablement les entreprises en fonction de leur situation. En outre, de nombreuses collectivités territoriales ont lancé des initiatives pour soutenir le tissu économique grâce à des aides spécifiques. Dans ce cadre, nous souhaiterions avoir des garanties sur la prise en compte, lors du contrôle de légalité, du caractère exceptionnel des difficultés Par ailleurs, nous saluons la décision de reporter d'un an les premiers remboursements des prêts garantis par l'État (PGE) ; c'est indispensable pour ne pas fragiliser davantage les entreprises déjà en difficulté. Une question subsiste toutefois sur les effets à long terme des PGE pour les entreprises qui, face à l'alourdissement de leurs dettes, seraient confrontées aux difficultés de remboursement et, plus largement, à des problèmes de liquidité.

de la Banque publique d'investissement, dont le renforcement des moyens d'investissement, dans un contexte de difficultés économiques pour les entreprises, est évidemment pour nous un motif de satisfaction,

manière plus spécifique, j'appelle, à titre personnel, l'État à prendre en compte l'ampleur de la crise économique et sociale en Corse, ainsi que la volonté unanimement exprimée par l'Assemblée de Corse d'y faire face de manière adaptée, en raison des conséquences majorées de la crise de la spécificité de notre tissu économique et social et de la structure de nos recettes fiscales, les circulaires de droit commun étant moins adaptées à la situation corse. Voilà les éléments que nous souhaitions porter à votre connaissance. Nous voterons bien sûr la ratification de ces ordonnances, que la menace d'un troisième confinement justifie d'autant plus. La parole

ce projet de loi de ratification est, pour nous tous, l'occasion de prendre un peu de recul par rapport aux mois interminables que nous venons de traverser. Cette situation exceptionnelle nous a conduits à confier au Gouvernement, comme la Constitution nous le permet, le soin de légiférer par ordonnances pour apporter une réponse massive à la crise. Le 12 mars dernier, le Président de la République annonçait la fermeture des établissements scolaires

La France entrait alors, aux côtés de ses voisins européens, dans une longue période d'incertitude, à laquelle se mêlaient les lointains échos de l'inquiétante rumeur qui commençait à nous parvenir de Chine, car nous ignorions encore tout de ce qui nous attendait. Tout s'est alors déroulé très vite. Dès le 18 mars suivant, le projet de loi d'urgence était transmis au Sénat et renvoyé à la commission des lois, tandis que la commission des finances de l'Assemblée nationale examinait le premier budget d'urgence le 19 mars, nous en terminions l'examen ; le 20 mars, le premier projet de loi de finances rectificative était adopté définitivement et, le 23 mars, les deux lois étaient promulguées. Il n'aura fallu que quelques jours pour élaborer et adopter ces deux textes et prendre des mesures d'une ampleur inédite, qui nous auront permis de faire face à la crise.

ont travaillé nuit et jour pour produire leurs précieux rapports, pour guider, conseiller et éclairer nos travaux, dans une période pourtant bien mouvementée. La brutalité de cette crise nous a conduits, je le disais, à habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances. Durant les trois premiers mois de l'épidémie, soixante-deux ordonnances ont été prises pour faire face à la crise et ont permis de soutenir les entreprises, les collectivités et l'ensemble des Français. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui en ratifie quatre. La première ordonnance qu'il nous est proposé de ratifier est l'ordonnance du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité. Ce dispositif, d'une ampleur sans précédent, aura versé, rappelons-le, plus de 12 milliards d'euros à près de 2 millions d'entreprises. Dans la Drôme, le département dont je suis élu, plus de 120 millions d'euros auront été distribués à 17 215 entreprises.

et de favoriser les PME, au même titre que l'ouverture des marchés de travaux sans publicité pour les lots de moins de 100 000 euros, adoptée lors de l'examen de la loi du La troisième ordonnance a permis de mettre en place la réorganisation de la Banque publique d'investissement, afin de permettre à cet établissement de déployer et d'administrer des prêts aux entreprises. La quatrième ordonnance, enfin, visait à faciliter l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté. C'est encore une mesure qui a permis d'apporter une réponse rapide et adaptée à la crise. la crise. Nous pouvons nous réjouir, je crois, d'avoir l'occasion d'examiner ces ordonnances et de les ratifier afin d'en sécuriser définitivement les dispositifs. Nous pouvons également nous féliciter de l'ampleur de la réponse de l'État et du Gouvernement pour faire face à ta crise. Pour ces deux raisons, le groupe RDPI votera ce texte.

-dans le contexte plus large du recours croissant aux ordonnances depuis une vingtaine d'années, principalement pour la transposition de directives européennes et pour l'application de textes en outre-mer, le plus souvent des sujets très techniques ou spécifiques. Le recours aux ordonnances avait été important sous le précédent quinquennat, avec l'état d'urgence lié aux attentats terroristes et la crise des frondeurs. Le gouvernement Philippe n'a pas été en reste, avec un nombre non négligeable de réformes adoptées par ce moyen, en particulier la réforme emblématique du code du travail en 2017-2018. L'année 2021 nous dira si cette tendance à la hausse se poursuit ou bien si nous allons revenir à un état plus « normal » des choses au regard de la procédure législative.

Cela pose la question du suivi et de l'exercice de la mission de contrôle des parlementaires : les ordonnances ont-elles bien été toutes ratifiées ? Le sont-elles toutes, habituellement ? Quelles sont les réelles marges de manoeuvre des parlementaires lors de l'habilitation et lors de la ratification ? C'est une discussion qui mériterait d'être approfondie, au-delà du texte que nous examinons aujourd'hui. Le présent projet de loi de ratification a été déposé dès le mois de juillet dernier, dans le respect des délais prévus dans la loi d'habilitation.

en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Je n'aurai rien de particulier à dire sur les différents articles. Il va de soi qu'il faut ratifier l'ordonnance du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées

-avait été succincte du fait de l'urgence et qu'il avait fallu attendre la publication du décret d'application, quelques jours plus tard, pour connaître les détails du fonctionnement de ce fonds, ce qui avait pu représenter des difficultés de compréhension pour les interlocuteurs de la société civile, au premier rang desquels se trouvaient bien sûr les entreprises. L'article 2, qui ratifie l'ordonnance du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique n'appelle pas davantage de commentaires. Des mesures exceptionnelles et relativement techniques ont été effectivement prises dans ce domaine, l'an dernier, afin de faire face à la suspension, voire à l'arrêt, des chantiers, surtout pendant le premier confinement, au printemps. L'article 3 ratifie une autre ordonnance datée du même jour, l'ordonnance du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement. Est ainsi opérée la fusion entre la société anonyme Bpifrance et sa filiale Bpifrance Financement, afin que le nouvel ensemble dispose de fonds propres plus importants, avec une participation publique qui reste très majoritaire. Les travaux de commission ont toutefois relevé que cette réorganisation amènerait à sortir la dette de Bpifrance du périmètre de la dette publique ; un élément supplémentaire à verser au débat qui grandit à ce sujet Enfin, l'article 4 ratifie une ordonnance relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté, dans le contexte de ralentissement économique actuel, avec des dérogations sur le plafond d'octroi des avances et le champ des bénéficiaires. Les députés ont adopté le présent projet de loi le 27 janvier dernier, avec quelques modifications qui vont dans le bon sens, en particulier la ratification de l'ensemble des dispositions relatives au fonds de solidarité prises

Cela dit, je prendrai le temps qui m'est accordé pour aborder le fonds de solidarité, la commande publique ainsi que la refonte de Bpifrance. Le Gouvernement a décidé de régler la crise sanitaire par ordonnances : soixante-deux

renforcer sa capacité à accorder des garanties ». Aujourd'hui, l'amorce d'un long processus de dépossession de la banque publique par les acteurs privés est à l'oeuvre, sans que nous puissions refuser l'accès des actionnaires à son conseil d'administration.

Le risque de non-remboursement des prêts garantis par l'État pourrait atteindre, selon Nicolas Dufourcq, directeur de Bpifrance, 7 % des souscripteurs. Ce scénario découle du faible taux de refus- 3 % -et représente un effet d'aubaine pour les acteurs bancaires, qui pourraient sortir de l'opération avec 2 milliards d'euros de bénéfice, quand l'État devra couvrir 8 milliards d'euros de pertes. Le volume de prêts accordés est deux fois moins important que ce qu'avait prévu le Gouvernement et 65 % des entreprises qui en ont bénéficié ne le décaisseront pas. pas. L'exclusion du champ des administrations publiques de la nouvelle BPI permet de s'affranchir des règles de déficit budgétaire, d'éviter le risque de contradiction avec le principe d'universalité budgétaire et de limiter l'autorisation du Parlement. Les crédits de la BPI risquent donc d'échapper au contrôle

ces services -, vous êtes dans l'obligation de recruter des contractuels pour pallier cette carence de personnel. Il est impératif de récupérer les 30 millions d'euros ciblés. Vous devez concilier contrôle et réactivité dans le versement des aides. Il y va du destin de nos entreprises fragilisées. La condition de la confiance retrouvée exige la garantie pendant plusieurs mois d'un montant minimum par catégorie d'entreprises. Notre amendement déclaré irrecevable allait dans ce sens, en prévoyant le versement d'un pourcentage de chiffres d'affaires perdu pour toutes les entreprises, loin de l'aide inéquitable de 1 500 euros, eu égard à leur situation économique.

La situation de crise que nous traversons l'exige : de manière transpartisane, nous devons nous montrer à la hauteur des difficultés auxquelles notre pays fait face. Ce n'est jamais de gaieté de coeur que nous acceptons de déléguer à l'exécutif notre précieux pouvoir de législateur, acquis acquis par nos illustres prédécesseurs dans les conditions que l'on sait, mais l'urgence de la situation nous y contraint. La première ordonnance prolonge l'existence du fonds de solidarité et renforce l'échange d'informations entre administrations. Il s'agit donc d'un outil incontournable pour soutenir notre tissu économique. Son rôle est essentiel pour les entreprises les plus en difficulté. La deuxième ordonnance comprend plusieurs dispositifs dérogeant temporairement au code de la commande publique. Elle introduit divers outils qui permettent de soutenir les opérateurs économiques les plus fragilisés par la crise. La troisième modifie l'organisation de Bpifrance, renforçant sa solidité financière, ce qui permettra des volumes de garantie de prêts plus importants. La Banque publique d'investissement va devoir jouer un rôle prépondérant dans le cadre du plan de relance. À ce titre, l'établissement public, en simplifiant sa structure, a fusionné sa holding de tête et sa filiale Bpifrance L'opération doit permettre d'augmenter le niveau des fonds propres et d'accroître sa capacité de financement des entreprises, mais nous ne sommes pas dupes sur le jeu d'écriture qu'implique une telle fusion.

Je note qu'un amendement présenté par le rapporteur tend à prendre en compte ce problème. Enfin, l'article 4 du projet de loi permet de ratifier l'ordonnance du 17 juin 2020 qui contribue à répondre aux besoins de trésorerie concomitants à la crise.

suivie de la crise des gilets jaunes, et, désormais, avec la crise sanitaire, nous constatons tous une sorte de recul des prérogatives du Parlement ou, du moins, une montée en puissance de pratiques gouvernementales basées sur le mépris ou,, un certain maintien à distance du Parlement, qui ne peut plus pleinement exercer correctement sa mission constitutionnelle. « La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude », cette habitude qui nous fait supporter le pouvoir d'un seul comme s'il était notre tout, cette habitude dans laquelle nous sommes plongés depuis un an au rythme des annonçant couvre-feu, confinement, déconfinement, nouveau couvre-feu, ... Qu'auriez-vous fait ? ... cette habitude qui rend si anxieux nos concitoyens ne sachant plus à quel saint se vouer. La Constitution de la V République permet au Président en place de prendre des décisions unilatéralement et de décréter que ses décisions personnelles sont l'intérêt commun. commun. Cela ruine la politique, au sens non pas partisan- il y a bel et bien une majorité et une opposition -, mais au sens de l'action publique, précisément comme bien commun. Mes chers collègues, comprenez-moi bien : je ne suis pas en train de dire raisonnablement à la tribune que le Gouvernement a failli dans sa prise de décision. Je tiens juste à souligner que les grands absents du processus décisionnel depuis le début de cette crise sont les élus du Parlement, ces élus remplacés par un conseil de défense qui se veut à la fois omniscient et omnipotent, qui décide de tout alors même que la composition de ses membres ne fait l'objet d'aucune onction démocratique.

Je m'étonne d'ailleurs que le Gouvernement n'ait pas directement transmis cette tâche au cabinet McKinsey, puisqu'il semble que ce soit dans l'air du temps ... Encore une fois, c'est non pas tant le phénomène que je dénonce- notre démocratie peut sans doute s'en accommoder -que son ampleur, dans une stratégie politique assumée qui vise à essayer de convaincre que, entre le Président sortant et le Rassemblement national, il n'y a pas d'alternative. La crise sanitaire a eu pour effet d'exacerber tous les maux de notre société que, jusqu'à présent, nous ne voulions voir. Notre système de gouvernance politique n'y a pas échappé. On le voit bien, le présidentialisme est au régime présidentiel ce que l'intégrisme est aux religions, ce que l'absolutisme est aux monarchies, ce que le sectarisme est aux convictions.

La situation sanitaire légitime le recours aux ordonnances, mais le fait que nous soyons amenés à légiférer dix mois après que le Gouvernement eut reçu l'autorisation d'écrire la loi et sept mois après qu'il l'eut effectivement écrite ne peut que nous interpeller. Ces délais démontrent, comme à l'accoutumée, l'indifférence profonde que vous portez au Parlement, lequel, dans votre esprit, semble se limiter à une caisse enregistreuse de décisions que vous avez déjà prises. Autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite », énonçait Ésope. Nous pensons que l'union devrait être plus forte entre le Gouvernement et le Parlement. Le pays y gagnerait, et c'est parce que nous ne voulons pas de défaite pour la France que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne s'opposera pas aux mesures que vous avez édictées de manière unilatérale. En conséquence, nous voterons favorablement ce texte, mais nous appelons l'attention de tous sur la situation critique qui est collectivement la nôtre et sur l'affaiblissement du Parlement que notre époque connaît. Il faudra rapidement revenir à un fonctionnement plus conforme à l'esprit de notre Constitution. Le parlementarisme rationalisé n'est pas un parlementarisme au rabais.

pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter celle-ci. Comme l'a rappelé notre rapporteur, soixante-deux ordonnances ont été publiées depuis. Le présent projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale le 27 janvier dernier, a pour objet de ratifier quatre d'entre elles, datant de juin 2020, afin d'en sécuriser juridiquement le dispositif. J'en resterai donc à ce cadre législatif et technique. L'article 1 tend ainsi à ratifier l'ordonnance du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Cette ordonnance a prorogé le fonds de solidarité jusqu'à la fin qui a permis de soutenir 2 millions d'entreprises l'année dernière, essentiellement des TPE et des PME, à hauteur de 13 milliards d'euros. Chacun mesure combien cela fut nécessaire. La ratification de l'ordonnance va permettre de ratifier le cadre juridique du fonds. L'article L'article 2 a quant à lui pour objet de ratifier l'ordonnance du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique. Cette ordonnance concerne les conditions d'accès aux marchés publics. Elle rend cet accès possible aux entreprises en redressement judiciaire qui bénéficient d'un plan de redressement. Cette mesure vise à soutenir les entreprises en difficulté du fait de la crise actuelle, qui n'auront plus besoin d'une habilitation. Il s'agit donc d'une mesure de simplification bienvenue dans le cadre de la relance économique, dont la commande publique constitue l'un des leviers importants. Cette relance doit aussi passer par la dimension territoriale. De ce point de vue, l'ordonnance va aussi permettre de privilégier les PME de proximité, en ouvrant aux petites et moyennes entreprises un accès privilégié aux marchés publics globaux, la fixation à 10 % de la part d'exécution minimale qui sera confiée par le soumissionnaire à des PME, et ce jusqu'au 31 juillet 2021. C'est essentiel pour nos entreprises. De surcroît, l'ordonnance prévoit que les critères d'accès aux marchés publics ne tiennent pas compte des conséquences, pour les entreprises, de la crise sanitaire. Ainsi, comme vous l'avez souligné, madame la secrétaire d'État, la baisse de chiffre d'affaires liée à l'épidémie ne pourra pas entrer en ligne de compte lors de l'examen par les acheteurs publics de la capacité économique d'une entreprise, cette baisse étant liée à un facteur externe. L'article 3 vise à ratifier l'ordonnance du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance du 29 juin 2005 relative à celle-ci. Cette ordonnance réorganise la BPI en fusionnant Bpifrance SA et sa filiale Bpifrance Financement, afin d'augmenter la solidité financière de l'ensemble pour pouvoir augmenter le volume de prêts accordés aux entreprises dans le contexte actuel. a permis, par exemple, de lever 400 millions d'euros lors du premier confinement, sans dotation de l'État supplémentaire, l'opération de réorganisation faisant plus que doubler le ratio de solvabilité de Bpifrance. Cette mesure avait été censurée comme cavalier dans le projet de loi ASAP. Pour le Gouvernement, il s'agit, en ratifiant l'ordonnance, de sécuriser juridiquement le dispositif. Enfin, l'article 4 prévoit la ratification de l'ordonnance du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque afin de renforcer le soutien financier apporté aux entreprises en difficulté dans le contexte de ralentissement économique actuel. Cette ordonnance permet des dérogations temporaires pour l'octroi de ces avances, qui sont un instrument important de renforcement des fonds propres des entreprises, en instaurant la possibilité d'impliquer le secteur privé en sus du secteur public. Les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque peuvent soutenir les entreprises touchées par la crise dont elles sont actionnaires au-delà du plafond légal habituel, correspondant à 15 % de leur actif. Ce plafond est, en effet, temporairement porté à 20 % jusqu'au 30 juin 2022. Au-delà, je pense que nous devrions ouvrir un débat sur les quasi-fonds propres des entreprises, en particulier sur le recours aux prêts participatifs, qui pourraient répondre à plusieurs enjeux afin d'assumer un effort d'investissement post-crise.

Personne ne pouvait alors imaginer que, un an plus tard, le bilan dépasserait 80 000 morts et que notre pays connaîtrait une récession sans précédent depuis 1945. Je me permets cette mise au point historique pour mieux rappeler la fulgurance avec laquelle le virus nous a frappés. Le 14 mars 2020, moins d'un mois après l'enregistrement du premier décès, le Gouvernement décidait de confiner le pays. Le 25 mars, une ordonnance était prise pour créer le fonds de solidarité et aider les petites entreprises face à la crise. Dans ce contexte, le Parlement a soutenu le Gouvernement en lui donnant la possibilité d'agir rapidement et efficacement par voie d'ordonnances. Ce n'est certainement pas la meilleure façon de légiférer en temps normal, mais c'est sans doute la meilleure manière d'agir avec la réactivité nécessaire en temps de crise. Voilà donc près d'un an que notre pays fait face à la pandémie. Loin de se résorber, celle-ci s'est installée dans la vie quotidienne et nous devons malheureusement encore aujourd'hui adapter nos réponses économiques à la crise sanitaire. C'est tout particulièrement le cas pour le fonds de solidarité. Depuis sa création, en mars dernier, les critères d'éligibilité, le niveau des aides dispensées et la pérennité de ce fonds n'ont cessé d'évoluer à mesure que notre pays s'enfonçait dans la crise. Mais sa vocation, elle, n'a pas changé. Je crois que nous pouvons tous attester de l'efficacité du dispositif dans nos territoires. Certes, les restaurants, les bars, les théâtres et tant d'autres établissements encore ne demandent qu'à rouvrir au plus vite. Mais tous saluent l'efficacité du fonds de solidarité, qui a été mis en place dans l'urgence et qui est progressivement monté en charge. C'est pourquoi il semble aujourd'hui tout à fait cohérent de poursuivre les efforts dans ce sens. La possibilité d'étendre la prise en charge à certains coûts fixes, en fonction des secteurs, pourrait aussi s'avérer pertinente dans les mois qui viennent. En tout état de cause, l'article 1 du projet de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans cette logique de réponse cohérente en soutien au tissu économique des territoires, singulièrement à nos artisans et à nos PME. L'article 2, bien qu'il ne concerne pas le fonds de solidarité, s'inscrit également dans cette logique de soutien aux entreprises des territoires, en activant un puissant levier d'action, à savoir la commande publique. Nous savons tous ici combien ce levier est important pour nombre de nos PME. C'est pourquoi les assouplissements prévus par l'article 2, qui vise notamment à permettre à des entreprises en redressement de se porter candidates et de mieux intégrer les PME dans les offres publiques, sont pertinents. D'ailleurs, le Sénat avait déjà adopté ces mesures lors de l'examen du projet de loi ASAP voilà un an. Je doute qu'il ait changé d'avis depuis, la crise n'ayant fait que renforcer la pertinence de ces mesures, qui n'ont jamais paru aussi salutaires qu'aujourd'hui. Avant de conclure, mes chers collègues, je souhaite dire un mot de la réforme de Bpifrance prévue par l'article 3. Je soutiens l'objectif affiché de renforcer ses fonds propres, afin de porter sa capacité de financement à 50 milliards d'euros d'ici à 2024. participe elle aussi à la cohérence de notre réponse économique à la crise sanitaire. Mais cette restructuration ne doit pas nous encourager sur le mauvais chemin de la dette. En effet, en faisant ainsi sortir la nouvelle structure faîtière des critères de Maastricht, nous soulageons artificiellement le fardeau de notre dette aux yeux de nos partenaires européens, avec lesquels nous avons pris, en responsabilité, des engagements de solidarité. Plus que jamais, le sort de nos finances publiques dépendra de la bonne santé de nos entreprises, qui ont contracté des prêts garantis par l'État, et du respect de nos engagements européens. Malgré ce point de vigilance, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte, qui constitue une nouvelle pierre au solide édifice de la relance.

la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant près d'un an est inédite, et les conséquences économiques qu'elle a entraînées sont considérables. Dans ces conditions, le Parlement a, dès le mois de mars 2020, été invité à habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances.

Certes, le projet de loi dont le Sénat est aujourd'hui saisi ratifie seulement quatre d'entre elles, mais il s'agit d'ordonnances importantes, relevant toutes du champ législatif des deux commissions des finances du Parlement. La première ordonnance, datée du 10 juin 2020, est relative au fonds de solidarité créé par l'ordonnance du 25 mars 2020, qu'elle a modifié et prorogé avant que la loi de finances pour 2021 ne le reconduise de nouveau. Le remaniement à diverses reprises de ce fonds aura permis d'ajuster les modalités de subventions suivant les secteurs, les catégories d'entreprises et l'impact économique subi, de façon à adapter le plus efficacement possible le soutien public à l'évolution et aux conséquences de la pandémie. la pandémie. Le fonds de solidarité a ainsi permis de soutenir à ce jour près de 2 millions d'entreprises parmi les plus touchées par la crise, représentant un engagement budgétaire de l'ordre de 15 milliards d'euros, dont 45 millions d'euros au bénéfice de plus de 6 200 entreprises de mon département du Jura. La réponse donnée par l'État fut rapide, diversifiée et massive : fonds de solidarité, chômage partiel, prêts garantis par l'État, report et sans doute, à terme, annulation au moins partielle des charges fiscales et sociales

sur l'éventuelle annulation des charges fiscales et sociales ? C'est une question cruciale pour toutes les entreprises bénéficiaires. Pour mener à bien le soutien, nous savons que les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) s'emploient sans relâche au déblocage rapide des aides que sollicitent les entreprises. Les contreparties à cette rapidité sont l'exigence et l'existence d'un contrôle rigoureux des bénéficiaires par l'administration fiscale, afin de traquer toute fraude. C'est ce que prévoit cette ordonnance, en offrant aux services fiscaux la possibilité de contrôler les bénéficiaires pendant une période de cinq ans. Nous nous en réjouissons. Nous nous félicitons de l'équilibre trouvé entre efficacité économique et équité sociale. La deuxième ordonnance, qui date du 10 juin 2020, assouplit opportunément les règles d'accès à la commande publique, essentiellement au bénéfice des PME. Certaines des dispositions qu'elle contient ont d'ores et déjà été inscrites dans le marbre législatif, à la faveur de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « ASAP ». Là encore, nous nous félicitons de ce que la crise ait été propice au pragmatisme et profitable à tous. La troisième ordonnance porte réorganisation de la Banque publique d'investissement. Cette réorganisation, qui a permis d'augmenter les fonds propres de Bpifrance, donc sa capacité de financement des entreprises, est, elle aussi, un motif de satisfaction pour les membres du groupe Union Centriste. Comme l'a rappelé notre collègue et rapporteur Bernard Delcros, que je tiens ici à saluer pour la qualité du travail effectué, la réorganisation de Bpifrance vise, au moyen d'une fusion-absorption de Bpifrance SA par l'établissement de crédit Bpifrance Financement, à surmonter le déséquilibre de la structure du point de vue de ses fonds propres. Outre la simplification de l'organisation et de la gouvernance de Bpifrance, cette réorganisation va permettre à l'établissement de crédit de bénéficier de la consolidation de Bpifrance Participations et, ainsi, de multiplier par plus de cinq le montant de ses fonds propres, qui devraient passer de 4 à 25 milliards d'euros, soit une augmentation de ses capacités à financer l'économie de l'ordre de 50 milliards d'euros d'ici à 2024. autre avantage significatif de la réorganisation concerne les modalités d'intervention de Bpifrance et leurs effets sur les comptes publics. La société de tête n'étant plus comptabilisée au sein des administrations publiques, Bpifrance pourra désormais, grâce à la garantie de l'État, s'endetter dans des conditions favorables sans que cela soit comptabilisé selon les critères de Maastricht. Les bénéfices de la réorganisation pour le soutien et la relance de notre économie seront immédiats, comme cela a été rappelé par notre rapporteur, un premier emprunt de 3 milliards d'euros est déjà prévu. Enfin, la quatrième ordonnance vise à faciliter l'octroi aux entreprises en difficulté d'avances de trésorerie en compte courant. Nous approuvons cette mesure, particulièrement bienvenue dans le contexte que nous connaissons. Elle participe pleinement aux réponses économiques qu'il nous faut apporter à l'épidémie de covid-19. Les membres du groupe Union Centriste se réjouissent aujourd'hui d'avoir l'occasion de débattre du contenu de ces ordonnances avant que leur soit conférée pleine valeur législative. Nous vous l'avons suffisamment rappelé, madame la secrétaire d'État : le Gouvernement ne doit pas exciper de la difficulté et de l'urgence de la situation pour contourner le Parlement et ses prérogatives. Nous avons ici été entendus et nous nous en félicitons, allant même jusqu'à espérer que la démarche sera prolongée dans les semaines et les mois à venir. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, notre groupe votera en faveur de cette ratification. La discussion

La raison est simple : il s'agit de redonner au tissu économique et associatif du pays les conditions pour sortir de l'incertitude liée à la crise sanitaire. Il y a un problème de conditionnalité de la stabilité des actions de l'exécutif national, madame la secrétaire

pour 2021. Il est encore temps de conditionner les aides du fonds de solidarité au maintien des salariés dans l'emploi. Il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures : on ne peut pas sanctionner des chômeurs et ne pas sanctionner les grandes entreprises qui ne tiennent pas leurs engagements.

il y a eu moins de défaillances en 2020 que les années précédentes. C'est logique : si vous fonctionnarisez tout le monde, il n'y a pas de défaillances ! Or c'est exactement ce qui a été fait.

notamment dans le domaine de l'innovation. Par ailleurs, Bpifrance et la Banque des territoires vont engager 40 milliards d'euros sur le plan Climat. Enfin, les investissements dans les entreprises stratégiques sont au coeur

: « Personne morale amorale, affectée d'un trouble oculaire spécifique : dans des comptes financiers, elle ne peut lire que la ligne du bas, celle du résultat. » Nous avons encore constaté cette amoralité des actionnaires avec le versement des dividendes en pleine crise sanitaire, malgré l'octroi d'aides publiques.

? La question du rôle de l'État actionnaire se pose au travers de cette incursion des acteurs privés. Nous sommes nombreux à fustiger le rôle de l'État dans le financement de l'économie ; nous le sommes un peu moins en temps de crise sanitaire- dont acte ! Reconnaissez tout de même que cette arrivée du privé est incohérente. Dès la création de la BPI, en 2012, qu'elle ne devait pas financer de « canards boiteux » ni rester dans les failles du marché pour laisser les activités les plus profitables aux acteurs privés. Ces derniers peuvent se rémunérer indirectement

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

pour 2021. Vous le savez, il existe différents moyens de financer cette activité de garantie. Il peut s'agir de crédits budgétaires, mais également de reprises de provisions ou d'utilisation des dividendes. L'opération de fusion n'apporte pas de changement sur ce plan. Il est en revanche plus que souhaitable que le Parlement puisse continuer de débattre en profondeur de l'avenir et des grands paramètres de l'activité de garantie de Bpifrance. Pour les exercices 2019 et 2020, alors qu'aucun crédit n'a été exécuté, l'activité de garantie de Bpifrance a bien été décrite dans les projets annuels de performance

ma chère collègue. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi est une réforme attendue par les courtiers et par les consommateurs. Nous avions eu l'occasion d'en débattre lors de l'examen de la loi Pacte, texte pour lequel

du Sénat. Comme présidente de la commission spéciale à l'Assemblée nationale sur la loi Pacte, j'avais à l'époque pleinement soutenu l'objectif de mieux accompagner les activités de courtage. Puis, le Conseil constitutionnel a finalement considéré l'article concerné comme un cavalier législatif. C'est un honneur d'être aujourd'hui devant vous, et peu de temps après le passage du texte à l'Assemblée nationale, pour réaffirmer notre désir commun en faveur d'une telle réforme. Ce texte apporte des réponses pragmatiques à nos entreprises de courtage pour pérenniser et renforcer la confiance des Français à leur égard, et donc leur viabilité. Il répond à la nécessité de protéger le consommateur, par la promotion d'un haut niveau d'exigence professionnelle pour l'ensemble du secteur. Au cours des dix dernières années, nous avons renforcé les règles en matière de protection du consommateur dans la sphère financière. Pourtant, force est de constater que ces règles ne sont pas toujours respectées : il y a, d'un côté, le manque de responsabilité de certains acteurs ; il y a aussi, de notre côté, parfois un manque de contrôle. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) n'est en mesure de réaliser que 70 contrôles par an, alors que nous avons près de 40 000 courtiers et mandataires en assurances et 13 000 courtiers et mandataires en opérations de banque et services de paiement. Au détriment de tous les professionnels de bonne foi, un tel contexte a permis le développement de pratiques malhonnêtes. Pour citer quelques exemples, nous pouvons parler du développement des garanties d'assurance construction placées chez des acteurs situés en dehors de nos frontières, à Gibraltar notamment. Faute de provisionnement adéquat, ces sociétés ont fait faillite en cascade à partir de la fin de l'année 2017, laissant les assurés sans aucune protection. Nous en avons tiré les leçons à l'échelon européen par un meilleur contrôle des activités transfrontalières. Mais nous devons aussi en tirer les leçons en France s'agissant de la distribution de garanties que l'on sait parfois douteuses. Je pense également à la pratique du démarchage téléphonique en assurance, qui s'est multipliée ces dernières années. La loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux était une première réponse. Je crois que nous pouvons aller plus loin pour contrer les purs schémas d'escroquerie et le démarchage abusif. J'aurai l'occasion de J'aurai l'occasion de vous présenter un amendement du Gouvernement en ce sens ; j'espère qu'il trouvera consensus ici. Pour que les Françaises et les Français puissent donner au courtage toute la confiance que ce métier mérite, il paraît indispensable que celui-ci s'organise, en actant la création d'associations professionnelles agréées, dont la relation avec l'ACPR sera consacrée dans la loi. Ces associations agréées seront chargées du suivi de l'activité et de l'accompagnement de leurs membres. À ce titre, elles offriront un service de médiation et vérifieront les conditions d'accès et d'exercice de l'activité, ainsi que le respect des exigences professionnelles, dans une logique de conseil et d'accompagnement. Dans le souci de favoriser la diversité nécessaire pour que chaque professionnel se sente à son aise, plusieurs associations seront créées. À ce jour, huit associations professionnelles ont déjà indiqué être prêtes à déposer leur dossier d'agrément. Cela démontre que le secteur est déjà en ordre de marche et, encore une fois, que cette réforme est attendue ou, en tout cas, trouve d'ores et déjà une réponse dans la pratique des professionnels. Les acteurs exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement pourront également adhérer à ces associations professionnelles agréées. Le droit européen ne nous permet pas de les y contraindre. Il s'agira donc d'une faculté, mais il est probable que la grande majorité de ces acteurs souhaiteront y recourir dès lors que cette adhésion constituera, pour les clients français, une marque de sérieux, d'engagement et un gage de confiance dans leur courtier. Concrètement, les associations agréées seront encadrées par des règles qui garantiront leur indépendance et leur impartialité. Quant aux professionnels, ils disposeront également de garanties importantes. Ainsi, la demande d'adhésion à l'association donnera lieu à une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. En cas de refus, celui-ci devra être strictement motivé et pourra faire l'objet d'un recours devant les tribunaux. En dehors d'une modification opérée en commission sur laquelle je vous proposerai de revenir un peu plus tard, le Gouvernement apporte aujourd'hui tout son soutien à cette proposition de loi nécessaire à la pérennité de notre réseau de courtage, en particulier des courtiers de proximité, dont la présence est si importante pour les assurés. les assurés. Nous souhaitons qu'elle puisse être promulguée dans les meilleurs délais, afin que sa mise en oeuvre puisse intervenir au printemps 2022 pour permettre une transition du secteur et renforcer dans la durée la présence des courtiers auprès des Français, en toute confiance. En cet après-midi,

nous examinons la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, introduite par notre collègue députée Valéria Faure-Muntian, sur laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée et qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Mon collègue Albéric de Montgolfier,

dans le cadre du projet de loi Pacte. Ce dispositif avait finalement été censuré comme cavalier par le Conseil constitutionnel. Sur le fond, la présente proposition de loi, examinée au sein de la commission des finances le 3 février, ambitionne d'organiser l'accès et l'exercice des professions de courtiers en assurances et en opérations de banque et en services de paiement. Les échanges que nous avons pu avoir en commission traduisent un constat clair : cette proposition de loi ne va pas révolutionner la profession de courtage en assurances et en services de paiement. Surtout, elle ne permettra pas de régler certaines difficultés majeures rencontrées par les courtiers et les consommateurs, sur lesquelles je reviendrai par la suite. Malgré tout, elle nous semble constituer un premier pas bienvenu, permettant d'accompagner les acteurs face aux défis réglementaires et commerciaux que doit relever la profession et de diffuser les bonnes pratiques au bénéfice des consommateurs. En effet, l'article unique de la présente proposition de loi prévoit la mise en place d'un système d'adhésion obligatoire à des associations professionnelles agréées par l'ACPR, qui seront principalement chargées d'accompagner ces professionnels, de fournir un service de médiation et de vérifier certaines conditions d'accès et d'exercice de leur activité. Ce système s'inspire de celui qui a été mis en place par la loi de sécurité financière de 2003 pour les conseillers en investissements financiers, financiers) dresse un bilan positif. Je précise que ces associations existent déjà et que six à huit d'entre elles devraient être agréées. L'entrée en vigueur de la réforme, initialement prévue pour le 1janvier 2021, a été reportée au 1 avril 2022 par nos collègues députés, pour tenir compte du décalage du calendrier lié à la crise. La mise en oeuvre de cette réforme est donc largement anticipée par les acteurs du secteur, et ce depuis la loi Pacte. Ils ne sont et ne seront donc pas pris au dépourvu. Les travaux de la commission des finances ont permis de faire évoluer le texte adopté par l'Assemblée nationale sur deux points essentiels. Tout d'abord, nous avons étendu les missions confiées à l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias), en prévoyant qu'il exerce le contrôle de l'honorabilité non seulement des dirigeants des structures concernées, mais également de leurs salariés : en clair, l'absence de condamnation pénale. Actuellement, l'Orias tient un registre des intermédiaires et dispose à ce titre d'un accès automatisé et sécurisé au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour vérifier les conditions d'honorabilité des seuls dirigeants. Dans sa première version, la proposition de loi aurait imposé aux associations agréées de demander les documents justifiant de l'honorabilité des dirigeants et salariés, ce qui aurait représenté une charge administrative non négligeable, pour un niveau de garantie plus faible. Il nous a donc semblé préférable de confier à l'Orias l'ensemble du contrôle des conditions d'honorabilité des dirigeants et salariés, dans la mesure où cet organisme dispose des habilitations et de processus de vérification déjà rodés. Le deuxième aménagement substantiel apporté lors de l'examen en commission concerne les domaines pour lesquels le droit européen interdit de confier aux associations des pouvoirs de contrôle, à savoir la fourniture de conseils, les pratiques de vente et la prévention des conflits d'intérêts. Pour ces derniers, nous avons permis aux associations agréées d'édicter des recommandations à l'égard de leurs membres. Cette évolution permettra aux associations de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et commerciales sans pour autant créer d'obligations pour leurs adhérents. étant, malgré les ambitions affichées par ses auteurs dans l'exposé des motifs, cette proposition de loi ne permettra pas de régler certaines problématiques pourtant majeures rencontrées par les courtiers et les consommateurs. D'une part, la proposition de loi n'apportera pas de solution aux dysfonctionnements de la libre prestation de services, qui s'est traduite- Mme la secrétaire d'État l'a rappelé -par des défaillances successives de plusieurs assureurs étrangers dont les polices étaient souscrites par des particuliers ou des professionnels en France, notamment- hélas ! -dans le domaine de l'assurance construction ou en automobile. En effet, le droit européen interdit de soumettre à une adhésion obligatoire les courtiers exerçants en France au titre de la libre prestation de service ou de la liberté d'établissement. D'autre part, la proposition de loi ne mettra pas fin aux pratiques commerciales déloyales parfois observées dans le secteur. En effet, les associations professionnelles ne seront pas habilitées à contrôler le respect des pratiques de vente et du devoir de conseil vis-à-vis des clients. Le système proposé diffère sur ce point de celui qui est en vigueur pour les conseillers en investissements financiers, qui peuvent être contrôlés à ce titre par l'association à laquelle ils adhèrent. Le règlement général de l'AMF impose même un contrôle sur place de chacun des membres au moins une fois tous les cinq ans. Il n'y a rien d'équivalent dans la proposition de loi, mais il s'agit, là encore, non d'un choix, mais d'une contrainte du droit européen, qui ne permet pas aux autorités publiques de déléguer leurs pouvoirs de contrôle dans ces domaines dans le champ de l'assurance. En dépit de ces deux limites, je pense qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. En effet, si les courtiers font l'objet d'un encadrement croissant à l'échelon européen avec la directive de 2016 sur la distribution d'assurances, les conditions d'exercice qui leur sont imposées sont peu contrôlées. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'ACPR réalise 70 contrôles par an, que 24 470 courtiers et 32 557 intermédiaires en opérations de banque et services de paiement sont immatriculés à l'Orias. Vous voyez le ...

les exigences d'accès à la profession sont souvent peu respectées. Avec le système proposé, les associations pourront désormais vérifier que les conditions d'exercice sont remplies, en particulier l'obligation d'offrir un service de médiation, de se former régulièrement et de souscrire à une garantie financière adéquate. C'est particulièrement nécessaire dans un secteur très atomisé où l'essentiel des acteurs- vous l'avez compris -sont des TPE. L'obligation d'adhésion devrait par ailleurs permettre de limiter le turnover et de décourager les projets professionnels les moins aboutis.

Il faut également garder à l'esprit que de nombreux intermédiaires ont déjà adhéré sur une base volontaire aux associations existantes et que la souscription comprend certains services, comme la médiation, auxquels les courtiers auraient de toute façon été tenus de souscrire. À plus long terme, la présence de plusieurs associations professionnelles nous paraît également de nature à susciter une modération de ces tarifs, dans une logique à la fois de concurrence et d'attractivité. Enfin, comme il ne s'agit pas d'embêter inutilement des professions déjà bien encadrées, soulignons que les agents généraux sont exclus du champ de l'obligation d'adhésion, y compris pour leurs activités accessoires de courtier. En effet, les assureurs opèrent une sélection stricte des candidats à l'exercice de la profession d'agent général, leur imposent des obligations de formation bien supérieures au minimum requis par le droit européen et les auditent régulièrement. Au total, et compte tenu des contraintes du droit européen, il nous semble donc que l'équilibre trouvé doit permettre de structurer la profession sans excès de zèle. C'est pourquoi la commission des finances vous invite à adopter cette proposition de loi. La parole

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui reprend un amendement porté par notre collègue Richard Yung et l'ensemble de notre groupe lors de l'examen de la loi Pacte, amendement qui avait également été soutenu par Jean Bizet et des membres de son groupe. Sénat l'avait alors très largement adopté, avec le plein soutien du rapporteur Michel Canevet et du Gouvernement. L'Assemblée nationale l'avait ensuite repris à l'identique, moyennant quelques aménagements rédactionnels. rédactionnels. Finalement, le Conseil constitutionnel, à l'issue de la navette parlementaire, avait choisi de le censurer comme « cavalier législatif ». C'est ainsi que nous nous retrouvons, deux ans plus tard, à examiner la proposition de loi de notre collègue députée Valéria Faure-Muntian, qui reprend cette disposition. Je ne doute pas qu'elle sera accueillie au Sénat avec le même enthousiasme qu'en 2019. Comme le rappelait Richard Yung dans son amendement initial, cette disposition tend à répondre à une situation qui n'a fait que s'aggraver au cours des dernières années et à laquelle il est urgent de remédier. Les marchés d'intermédiation bancaire et assurantielle se sont fortement développés dans un contexte historique de taux bas et d'essor de l'offre de produits financiers. Le contrôle exercé sur cette offre est assuré par l'ACPR, mais n'est plus tout à fait adapté à ces nouvelles structures et à un marché d'intermédiation de plus en plus éclaté. C'est pour cette raison que la proposition de loi écarte l'option d'une surveillance directe par l'ACPR, pour confier cette mission à des associations agréées. En effet, l'ACPR réalise un peu moins d'une centaine de contrôles par an, face à un marché de près de 13 000 courtiers et mandataires en opérations bancaires et services de paiement et de plus de 40 000 courtiers en assurances. L'ACPR n'est manifestement pas en mesure d'assurer seule l'encadrement du secteur du courtage. Cette proposition de loi présente donc une solution équilibrée qui prend exemple sur le dispositif existant pour les conseillers en investissements financiers, fondé sur l'intervention d'associations agréées et qui permet un contrôle efficace du secteur. Les associations agréées auront un rôle complémentaire de ceux de l'ACPR et de l'Orias. Il ne s'agit nullement de retirer des compétences à ces organismes, comme certains semblent s'en inquiéter, mais au contraire de les seconder et de les renforcer. J'aimerais ici reprendre un exemple qui avait été cité lors de l'examen de la loi Pacte et qui se produit malheureusement encore trop souvent, celui d'un client de bonne foi qui aurait souscrit une assurance construction auprès d'un courtier installé en France. lorsqu'il souhaite déclarer un sinistre et faire jouer son assurance, la société, curieusement domiciliée à Chypre, Malte ou Gibraltar, a disparu et n'est plus là pour honorer son engagement. Nous le voyons bien, il est urgent d'améliorer les conditions de commercialisation des produits d'assurance et de services bancaires et il est essentiel de responsabiliser les courtiers sur les produits qu'ils vendent. C'est au fond l'objectif de l'amendement n° 2 du Gouvernement, qui tend à mieux encadrer les démarchages téléphoniques et à interdire les ventes « en un temps », qui se transforment encore trop souvent en escroqueries visant les personnes âgées ou les plus vulnérables.

C'est une excellente réponse à ceux qui demandent de retarder de nouveau l'entrée en vigueur de la proposition de loi. Cette réforme est attendue par les professionnels et par les consommateurs. La date du 1 janvier 2022 prévue pour son entrée en vigueur me semble être un bon compromis entre le temps qu'il faudra laisser aux acteurs pour s'adapter à la nouvelle réglementation et la nécessité d'encadrer au plus vite les mauvaises pratiques de certains. J'aimerais enfin répondre à ceux qui relevaient à juste titre en commission que les acteurs étrangers exerçant des activités en France ne seraient pas obligatoirement soumis à ces nouvelles obligations, en raison d'un droit européen qui ne permet pas de les y contraindre. Il ne faut pas oublier l'effet d'entraînement d'une telle mesure sur l'ensemble du secteur, car l'adhésion à une association agréée constituera pour les clients français un gage de fiabilité. C'est un cercle vertueux qui permettra d'assainir peu à peu le marché et de rétablir la confiance en responsabilisant les acteurs. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI soutiendra cette proposition de loi.

Il désigne un intermédiaire des échanges chargé de la mise en relation, ou encore de l'entremise d'un vendeur et d'un acheteur potentiels. Le mot « courtier » trouve ses origines dans l'occitan « corratier » ; c'est un coureur ou une personne qui court pour réaliser des opérations commerciales. On le trouve au Moyen Âge sur les marchés ou dans les ports. Outre le fait qu'il doit avoir de bonnes jambes, le courtier doit aussi savoir créer et entretenir d'excellentes relations avec les différentes parties concernées. Parfaitement informé, il sait qui vend et qui souhaite acheter. À cette époque, chaque courtier avait sa spécialité propre. Dans mon département, le courtier en vin était un personnage particulièrement important. En finances, le courtier peut être un intermédiaire qui agit soit sur les marchés financiers pour le compte de tiers, soit en mettant en relation deux parties avec pour objectif qu'elles contractent ensemble. Le courtage est devenu une activité très présente en bourse et dans les activités financières en général, mais il a fortement décliné ou s'est transformé, ces dernières années, avec l'automatisation du et la numérisation. Aujourd'hui, il se développe particulièrement dans le domaine des brevets, de la propriété intellectuelle et le commerce des données, sans oublier, de façon plus anecdotique, le courtage matrimonial L'objet de cette proposition de loi, repris d'une disposition censurée de la loi Pacte de 2019, est plus restreint, dans la mesure où il porte sur le courtage dans le domaine des assurances et des opérations de banque. Sur le fond, il y a peu de choses à ajouter à ce qui a été dit. Le texte a déjà été amendé à l'Assemblée nationale et lors de l'examen en commission. La volonté du Gouvernement de faire avancer ce sujet semble intacte, malgré la situation économique fortement bouleversée depuis un an par la pandémie. Il est vrai que cette réforme devait initialement entrer en vigueur au 1 janvier ... On peut regretter certains « angles morts » de la proposition de loi, comme le courtage en immobilier, secteur différent il est vrai, mais qui intéresse nos concitoyens. Si ce texte n'est pas un texte « fourre-tout », le terme de courtage lui-même reste très large, car il y a autant de métiers et d'intermédiaires que d'activités commerciales. L'application stricte de l'article 45 de la Constitution réduit l'initiative parlementaire à des ajustements techniques, là où il y aurait matière à mieux encadrer un certain nombre d'activités qui relèvent du courtage. Je salue néanmoins les avancées présentes et remarque que le texte recouvre bien des activités telles que le courtage en crédit immobilier. Les courtiers en opérations de banque répondent au terme de « IOBSP »- intermédiaires en opérations de banque et services de paiement. Comme les courtiers en assurances, ils apparaissent très nombreux ... On peut attendre de l'adoption du présent texte que ces secteurs s'organisent davantage, du fait de la nécessité d'effectuer des démarches supplémentaires d'agrément. Cela devrait avoir un effet bénéfique pour le consommateur, dans le respect des règles de juste concurrence. L'obligation d'adhésion à des associations professionnelles agréées par l'ACPR permettra, espérons-le, un meilleur contrôle, tout en conservant un système souple et la liberté d'établissement et de services. Son objectif, présenté lors des débats sur la loi Pacte, est avant tout de lutter contre certains abus, comme dans la vente de contrats d'assurance construction ou automobile, où des clients ont pu être abusés par des sociétés frauduleuses parfois domiciliées à l'étranger. L'examen à l'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications ou de précisions. Les refus d'adhésion par les associations devront être motivés, et les professionnels bénéficieront de moyens de recours. À l'inverse, les associations agréées pourront informer les autres associations d'un retrait de la qualité de membre. Surtout, l'entrée en vigueur est décalée au printemps 2022 du fait de la crise sanitaire, avant la fin du quinquennat

les limites intrinsèques du texte, qui doit respecter le cadre défini au niveau européen par la directive sur la distribution d'assurances de 2016, dite « DDA laquelle interdit une coopération trop poussée entre les pouvoirs publics et les représentants du secteur, au nom de la liberté de service et de la non-interférence avec les autorités étrangères homologues.

je vous remercie Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « il existe des contrats pour vous protéger contre toutes les calamités imaginables, sauf contre les démarcheurs de compagnies d'assurances ». Ce proverbe populaire pointe le paradoxe que propose de résoudre cette proposition de loi.

Le grand public avait découvert leur existence au moment du scandale qui avait éclaté dans le secteur de l'assurance construction. Des dizaines de milliers d'assurés, qui avaient souscrit des assurances des courtiers grossistes auprès d'assureurs exerçant en LPS, se sont retrouvés bien démunis lorsque leurs problèmes ont commencé. Les pratiques frauduleuses des LPS sont désormais bien connues : concurrence déloyale sur les prix et faillite lorsqu'il faut payer les sinistres. La problématique est malheureusement diffuse. La spécificité des contrats dits « décennaux fait peser pendant dix ans le risque de s'exposer aux pratiques frauduleuses de certaines compagnies d'assurances parfois établies dans des paradis fiscaux. Le cas de Gibraltar en est un exemple : on compte une entreprise d'assurance pour 700 habitants dans ce paradis fiscal, contre une pour 220 000 en France. L'auteure et rapporteure du texte à l'Assemblée nationale reconnaît que les assureurs en LPS constituent « un problème très complexe et sensible ». Pourtant, ce texte ne résoudra pas la problématique des acteurs en libre prestation de services en difficultés financières ou même en faillite, dont les contrats demeurent distribués par des courtiers français.

Cette proposition de loi risque finalement de subir le même sort que la disposition contenue dans la loi Pacte, en s'exposant, non pas à une censure du Conseil constitutionnel cette fois, mais à une contestation au motif de sa non-compatibilité avec le droit européen.

qui doivent être exercées par « des autorités publiques » ou « des organismes reconnus par le droit national », et non par « des associations dont les membres comprennent directement ou indirectement des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance

n'épargne pas les syndicats professionnels, qui se chargent d'ores et déjà de la veille juridique, de faciliter la formation professionnelle et d'assurer des missions de médiation par l'entremise de la « médiation de l'assurance ». Ce sont d'ailleurs ces mêmes syndicats professionnels qui créeront les associations agréées dont il est question dans cette proposition de loi.

En creux se dessine le risque que le dialogue social de la branche professionnelle se délite et que le Gouvernement dispose des coudées franches pour imposer ses vues au secteur. Les associations agréées ne joueront pas non plus ce rôle de dialogue, car elles seront atomisées. Il pourrait en exister entre quatre et six. Quel est le fondement d'une telle concurrence ? L'adhésion étant obligatoire, un acteur unique nous paraissait plus adapté, d'autant que les associations seront amenées à délivrer des recommandations. Celles-ci formuleront pour les mêmes acteurs de l'assurance des conseils différents. Leur portée, au-delà d'ajouter de la confusion, sera donc nulle. Je ne reviens pas sur les risques de conflit d'intérêts de l'auteure de la proposition de loi, qui ont été mis en lumière par Mediapart. Même si elle déclare ne pas s'être posé de questions « sur le coup » à propos de son lien avec le Intermedius, elle a changé d'avis en déclarant après le dépôt du texte un lien d'intérêt bénévole avec la structure. Enfin, il est tout de même curieux de constater que ce texte, pourtant construit par les acteurs du secteur, ne contente au fond pas pas grand monde. Pour les sénateurs et les sénatrices du groupe CRCE, nul besoin d'ajouter une strate inutile, qui, contrairement à l'objectif affiché, n'améliorera pas la protection du consommateur. La parole

présentée par notre homologue députée de la Loire Valéria Faure-Muntian, la proposition de loi que nous examinons vise à réguler et à structurer les activités de courtage en assurances et en opérations de banque et services de paiement. Ce texte entend non seulement accompagner les professionnels d'un secteur aujourd'hui largement éclaté, mais également garantir aux consommateurs une meilleure protection, en renforçant un cadre juridique jugé trop évasif. Le dispositif qui nous est proposé dans ce texte reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 207 du projet de loi Pacte, que le Conseil constitutionnel avait censurées au motif qu'il s'agissait de cavaliers législatifs. nous accorderons tous sur ce constat : le droit en vigueur n'offre pas de cadre suffisant aux métiers de courtier en assurances et d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Or l'expansion du marché et, à travers elle, la nécessité d'un meilleur contrôle des exigences professionnelles requises invitaient le législateur à se saisir du sujet à bras-le-corps. Les marchés d'intermédiation bancaire et assurantielle ont en effet connu une forte croissance ces dix dernières années. Depuis 2010, le nombre de courtiers en assurances a ainsi progressé de 25 %. Celui d'intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement a, quant à lui, bondi de 60 % depuis 2016. Cette augmentation exponentielle s'explique de différentes façons. Elle tient tout à la fois aux habitudes nouvelles prises par les consommateurs, à la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne et aux nouveaux produits d'épargne mis en place à la faveur de la loi Pacte. L'activité de courtage s'est en somme développée plus rapidement qu'elle ne s'est organisée et professionnalisée. Afin d'y remédier, la présente proposition de loi s'inspire directement du modèle de corégulation appliqué aux conseillers en investissements financiers, lequel est fondé sur une obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers. Très concrètement, aussi bien pour les courtiers d'assurance ou de réassurance que leurs mandataires et les intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement, le texte prévoit d'instaurer l'autorégulation des secteurs d'intermédiation bancaire et assurantielle, en s'appuyant sur une adhésion obligatoire à des associations professionnelles, agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Deux raisons principales conduisent le groupe Union Centriste à soutenir l'esprit et le contenu de la proposition de loi qui nous est ici soumise. Tout d'abord, l'accompagnement des intermédiaires de l'assurance et des services bancaires, qui, pour la grande majorité, sont des TPE, se voit opportunément renforcé. Ces intermédiaires trouveront désormais des interlocuteurs fiables au sein de ces associations pour les conseiller, afin qu'ils se conforment aux évolutions du cadre réglementaire de leur profession. Nous nous en réjouissons. le choix d'une assurance ou de services bancaires est un moment important dans la vie de nos concitoyens et des consommateurs, qui peuvent à cette occasion s'engager pour de très longues années dans un plan de remboursement. Il est donc de notre devoir de leur garantir une protection nécessaire, ce que prévoit le présent texte. Là aussi, nous nous en félicitons. Le groupe Union Centriste n'en est pas moins sensible aux lacunes soulevées par le rapporteur, Albéric de Montgolfier, dont nous voulons saluer le travail accompli au nom de la commission des finances. Nous pouvons en effet regretter que le dispositif ne soit pas en parfaite adéquation avec les ambitions affichées par les auteurs de la proposition de loi. Certes, ce décalage ne leur est pas entièrement imputable, les insuffisances du texte, en particulier quant au contrôle des conditions de commercialisation des produits d'assurance, tenant- cela a été rappelé à plusieurs reprises -aux fortes contraintes du droit européen qui pèsent sur notre législation nationale. Ainsi la réglementation européenne empêche-t-elle de soumettre à une adhésion obligatoire les intermédiaires étrangers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement, un écueil qui, hélas, risque de poser de sérieux problèmes d'équité De même la réglementation européenne empêche-t-elle rigoureusement de transposer aux courtiers en assurances et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement le modèle de corégulation qui existe pour les CIF. Là encore, cela constitue un obstacle préjudiciable et une limite au texte que nous examinons.

d'autant plus vrai que le dispositif issu du texte transmis par l'Assemblée nationale a pu être substantiellement enrichi par la commission des finances du Sénat. Le transfert du contrôle de l'honorabilité des dirigeants et des salariés à l'Orias, de même que la faculté offerte aux associations professionnelles d'émettre des recommandations vis-à-vis de leurs membres en matière de pratiques commerciales et professionnelles vont ainsi dans le bon sens Vous l'aurez donc compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste soutiendra cette proposition de loi. La parole

la proposition de loi que nous examinons a pour objectif d'organiser l'autorégulation des professionnels du courtage en assurances. Elle intervient à la suite de la censure de la loi Pacte par le Conseil constitutionnel, qui avait vu, à l'époque, dans les dispositions reprises par ce texte des cavaliers législatifs. En ce sens, je le note, nous avons affaire à un projet de loi sous forme de proposition de loi. De ce fait, nous ne disposons pas d'une étude d'impact à proprement parler. Le secteur du courtage compte de très nombreux acteurs et connaît un très fort turnover. Des scandales récents ont révélé la nécessité de le réguler davantage dans le but de remédier aux dysfonctionnements réglementaires constatés et, ainsi, de mieux protéger les consommateurs. Ce texte très technique, ramassé en un seul article, souhaite donc structurer ce secteur autour d'associations professionnelles agréées à adhésion obligatoire.

Cette réforme de la profession du courtage concerne près de 56 000 professionnels, lesquels sont soumis aujourd'hui à un premier autocontrôle du fait de leur enregistrement au registre de l'Orias, cet enregistrement étant nécessaire pour exercer. Un second contrôle peut intervenir de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, chargée de vérifier la véracité des documents transmis à l'Orias et les pratiques des courtiers. À ce titre, l'ACPR a encore récemment sanctionné un courtier pour des manquements en matière de démarchage commercial. Pour mémoire, ces organismes ont été mis en place à la suite de la crise financière de 2008 afin de garantir les services assurantiels. Les contrôles effectués par l'ACPR sont trop peu nombreux : seulement 70 en 2020. Cette proposition de loi entend donc y remédier. Pourtant, malgré les bonnes intentions des auteurs, le contenu du texte est décevant et loin des ambitions formulées dans l'exposé des motifs. Alors qu'il nous est présenté comme un renforcement des garanties pour le consommateur, dans les faits, ce texte consiste en la création d'associations de contrôle. D'une part, ce texte n'apportera pas de solution aux dysfonctionnements de la libre prestation de services, alors même que de nombreuses défaillances ont été relevées dans le secteur du bâtiment et de l'assurance automobile. De même, rien n'est précisé quant au devoir de conseil vis-à-vis des clients. D'autre part, c'est une manière pour l'autorité de régulation de déléguer sa mission de contrôle à des acteurs privés ayant leurs propres règlements. C'est donc une régulation de marché et en même temps un recul de l'État

favorisant de fait les grosses entreprises de courtage. Elle organise donc une dérive oligopolistique sur un marché qui n'en a pas nécessairement besoin, et cela au détriment des consommateurs. Contrairement à l'intention présentée par les auteurs, concentrer de la sorte les acteurs sur le marché mènerait à pousser les prix à la hausse par le mécanisme d'offre et de demande. Enfin, cette réforme génère une surlégislation en créant un intermédiaire supplémentaire entre les professionnels et les instances nationales de régulation. mes chers collègues, mon scepticisme quand, lors du PLF, on supprime l'obligation d'adhésion à des organismes de gestion agréés, qui jouent un rôle similaire sur un autre marché, avant d'adopter quelques semaines plus tard la logique parfaitement inverse avec ce texte. avec ce texte. Une simple réforme réglementaire aurait pu permettre d'augmenter la fréquence des contrôles de l'ACPR. En effet, avec près de 6 millions d'euros de cotisations récoltées, elle devrait avoir les moyens de se consacrer à ces contrôles. aurait-il été opportun d'examiner la situation d'un peu plus près avant de déléguer purement et simplement ses missions à des associations agréées. De même, afin de protéger davantage les consommateurs, il serait nécessaire que les courtiers aient recours à des services de médiation. Pour les y inciter, un justificatif mentionnant ces services pourrait être exigé lors du renouvellement de l'inscription au registre de l'Orias. Autre point important cette réforme souligne également les besoins de formation continue et d'accompagnement. Cette problématique dépasse largement le secteur bancaire et assurantiel et nécessiterait une réflexion plus large. Pour autant, en l'espèce, l'Orias pourrait, là encore, demander aux intermédiaires, au titre de la formation continue, tout document attestant des formations suivies et de la qualité de celles-ci. Avant de conclure, j'ajouterai deux remarques de méthode sur cette réforme. En premier lieu, je regrette, comme je l'ai déjà dit, l'absence d'une étude d'impact qui aurait éclairé ce texte très technique. Une telle étude aurait pu démontrer pour quelles raisons nous devrions organiser un marché plus concentré et en quoi cette organisation aurait pu être favorable aux consommateurs. En effet, malgré la volonté affichée de protection des consommateurs, il n'y a rien dans ce texte qui garantisse une augmentation des droits ou la possibilité d'un recours. lieu, au regard de la crise sociale inédite que nous traversons, le groupe socialiste ne comprend pas l'urgence d'une lecture de cette proposition de loi en procédure accélérée et sur le temps gouvernemental. Il y a effectivement de vraies urgences à traiter dans notre pays. Elles sont sanitaires, sociales et environnementales. Par ailleurs, ce texte de loi ne mérite pas d'être travaillé dans l'empressement d'un calendrier contraint par les échéances électorales à venir. Ces dispositions, qui entendent réguler un secteur d'activité, désarment en fait la puissance publique au lieu de lui donner les moyens d'exercer ses missions et d'effectuer les contrôles qui seraient nécessaires à la réelle protection des consommateurs. Ces derniers sont quand même les laissés-pour-compte de ce texte alors qu'ils en étaient la principale justification. Cependant, au-delà de la méthode qui n'est pas la bonne et ne permettra pas d'être efficace, ce texte a le mérite d'engager la réflexion sur une problématique réelle. Nous serons à cet égard très attentifs quant à la traduction réglementaire de ce texte de loi une fois son adoption actée. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe socialiste s'abstiendra sur ce texte, qui n'apporte pas de solutions en matière de protection des consommateurs.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, sous des aspects très techniques, le texte que nous examinons aujourd'hui renvoie à une réalité bien connue de nos concitoyens quiconque a déjà souhaité comparer différentes offres d'assurance ou de prêt a éprouvé le besoin d'être aidé dans ses démarches. C'est justement le rôle du courtier que d'apporter cette aide. Le courtage opère comme un intermédiaire entre l'assureur ou la banque, d'une part, et le client, d'autre part. Son rôle consiste à agréger différentes offres de prestation afin de faire jouer la concurrence et d'apporter les solutions les mieux adaptées aux besoins des clients. Comme pour toute offre d'intermédiation entre le fournisseur d'une prestation et son bénéficiaire, le courtier crée de la valeur quand il génère de la confiance entre l'un et l'autre. Il s'agit de trouver, pour le client, l'offre la mieux adaptée et au meilleur prix. Aujourd'hui, cette profession regroupe des acteurs très nombreux et très divers. Sont ainsi immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance 25 000 courtiers en assurances, 34 000 intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et près de 7 700 entreprises étrangères intervenant en prestation de services ou en libre établissement sur le sol français. Il est utile de rappeler ces chiffres, car ils illustrent bien la réalité du marché du courtage en assurances et en opérations de banque. Ainsi, lorsqu'ils cherchent à souscrire une police d'assurance ou s'apprêtent à s'engager dans un crédit, les consommateurs font face à une myriade d'acteurs qui n'ont ni les mêmes statuts ni les mêmes exigences en matière de transparence.

existe à cause de certains, c'est l'ensemble des acteurs qui en font les frais et, au bout de la chaîne, le consommateur. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants soutient le principe de cette démarche de réforme : il apparaît judicieux de renforcer les contrôles prudentiels réalisés sur les entreprises. La création d'associations professionnelles à adhésion obligatoire, soumises à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, doit permettre de rendre l'offre de courtage plus lisible et plus transparente pour les consommateurs. J'ai entendu les arguments selon lesquels l'entrée en vigueur de ce dispositif était précipitée. C'est vrai que la date, fixée par l'Assemblée nationale au 1 avril 2022, ne laisse guère plus d'un an aux acteurs et aux nouvelles associations professionnelles pour s'organiser. Mais cet argument omet le fait que les concertations ont été engagées dès 2018 et que le Parlement avait déjà voté cette réforme dans le cadre du projet de loi Pacte avant que le Conseil constitutionnel ne supprime les articles concernés au motif qu'ils constituaient des cavaliers législatifs. Je pense que nous devons avant tout veiller à ce que cette réorganisation de la profession ne fasse pas peser sur les acteurs économiques, par le biais des cotisations d'adhésion, des surcoûts qui seraient répercutés sur les consommateurs. Mis à part ce point de vigilance, notre groupe soutient cette réforme,

Dès lors, la seule question qui vaille en réalité est de savoir si ce texte y concourt vraiment. Permettez-nous d'en douter au regard des nombreuses questions que soulève ce texte. Tout d'abord, rappelons que, d'inspiration gouvernementale, cette proposition de loi issue de la majorité à l'Assemblée nationale s'apparente- disons-le clairement -à un projet de loi qui ne dit pas son nom. Preuve de cette ambiguïté à peine cachée, l'oubli initial du gage pour la charge supplémentaire créée par la nouvelle compétence d'agrément des associations par l'ACPR. Ensuite, le texte fait l'économie d'une étude d'impact qui aurait sans doute été utile pour apprécier le dispositif proposé, dont le fonctionnement reste ardu et que vous nous demandez de voter presque à l'aveugle. En outre, nous nous interrogeons sur l'articulation du texte avec le droit européen. Si la directive de 2016 prévoit bien que des courtiers peuvent fonder des associations de cadrage, il reste que les activités de contrôle doivent être réservées à l'autorité publique.

n'aurait-on pas eu plus intérêt à étudier la possibilité de renforcer les moyens de l'ACPR pour qu'elle puisse suivre l'évolution du secteur ? Par ailleurs, nous nous interrogeons sur les modalités d'application de la réforme : elles doivent être précisées par décrets en Conseil d'État, c'est-à-dire sans aucune intervention du Parlement. En l'absence d'étude d'impact, ce texte pose problème. Les gagnantes semblent être les associations professionnelles, qui bénéficieront de cotisations, sans que rien assure l'efficacité de l'autorégulation évoquée. L'adhésion obligatoire des courtiers constitue pour lesdites associations une manne financière considérable. Elles sont de fait en situation de conflit d'intérêts : en excluant un de leurs membres, elles perdront leur cotisation. Dès lors, quelle sera leur motivation réelle à agir en faveur de l'autorégulation ? Pire encore, ces associations professionnelles au service des courtiers pourraient devenir des groupes d'intérêts et aggraver le problème initial de régulation. N'aurait-il pas été préférable de taxer les banques, les assurances et les courtiers à hauteur à hauteur de leurs dépenses consacrées à la mise en conformité aux règles prudentielles afin de financer un contrôle externe et renforcer les moyens de l'ACPR et de l'AMF condition, la puissance publique aurait peut-être pu s'assurer que certains ne profitaient pas de l'aubaine constituée par un désert juridique et un encadrement assez évasif. Dès lors, ce texte, certes amélioré en commission, semble répondre partiellement aux objectifs, pourtant louables, que ses auteurs mais au risque de me répéter, il est impossible, en l'absence d'étude d'impact, d'évaluer les effets de cette réforme. Il nous semblait que, au regard de la crise que traverse la France et des terribles difficultés qu'endurent les citoyens, la mise en place de dispositifs de soutien à leur égard était plus prioritaire. Aussi aurions-nous largement préféré discuter de la place que prennent les assurances dans le soutien à la population, alors que le contexte sanitaire, économique et social extrêmement préoccupant exige une mobilisation sans faille du Parlement. C'est donc au regard du droit du Parlement à légiférer dans des conditions acceptables et de ne pas être réduits à une fonction d'approbation, mais également, car aucun élément n'accrédite l'idée d'une meilleure protection du consommateur,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que nous devions marcher vers une simplification massive de l'administration, alors que nous ne cessons de dénoncer, comme une majorité de Français, le poids de la suradministration, des normes et des régulations dans tous les domaines, comme la santé ou la recherche, et alors que

pas loin de 11 000 chaque année. J'ai également pris conscience que les courtiers en assurances devaient remplir des obligations de médiation, de formation et de garanties financières. Cet aspect est aujourd'hui peu suivi compte tenu de la taille moyenne des structures.

Dans le texte que nous examinons aujourd'hui, il est proposé que les courtiers en assurances qui dépendent de l'autorité de contrôle, à savoir l'ACPR, et sont immatriculés à l'Orias dès leur installation et dont l'adhésion est renouvelée chaque année soient adhérents d'une association professionnelle à partir du 1 avril 2022.

Le contrôle et la sanction des mauvaises pratiques resteront à la charge de l'ACPR, et l'Orias poursuivra ses missions sans étendre ses compétences. Ces associations auront la possibilité de prévenir l'ACPR et les autres associations en cas d'irrégularité,

Le risque, c'est bien qu'à nouveau la libre concurrence et la recherche d'innovation fassent les frais de ce formalisme normatif contraignant. Il est indispensable pour un assuré de pouvoir juger lui-même de la compétence d'un courtier motivé par le mérite et la passion. L'uniformisation des pratiques serait contraire à l'intérêt de l'assuré. Le Gouvernement s'était d'ailleurs engagé à défendre la liberté d'entreprendre et d'innover, mais quelle ne fut pas ma surprise en voyant l'amendement qu'il a déposé en dernière minute et qui a pour but d'imposer à tout intermédiaire en assurances d'enregistrer ses conversations téléphoniques avec ses clients et de les archiver pendant deux ans, le but étant prétendument de limiter le démarchage commercial des plateformes d'appel. L'idée est louable, si c'est pour éviter le démarchage commercial par des plateformes à distance qui ne respectent pas la vulnérabilité des personnes, mais mais l'amendement reste compliqué à accepter pour les professionnels, assureurs et banquiers, qui ne pourront appeler un prospect ou un client pour lui faire une nouvelle offre sans enregistrer la conversation.

fait, vous ne réglerez pas le problème réel, mais vous handicaperez des professionnels de proximité qui travaillent sur l'ensemble du territoire. Je regrette que cet amendement ait été déposé sans concertation avec les professionnels de l'assurance et de la banque. La commission des finances a d'ailleurs déposé un sous-amendement afin que cette disposition soit revue avec les professionnels et mieux adaptée à l'objectif. En conclusion, je dirai que cette proposition de loi impose à nouveau un coût non productif aux courtiers en assurances du territoire, sans régler le problème de la concurrence étrangère peu scrupuleuse.

des garanties inutiles. Ces pratiques sont minoritaires, mais elles sont en réalité un fléau pour tout le monde et nuisent considérablement à la crédibilité du secteur. La disposition qui vous est proposée ici fait l'objet d'un consensus de place

amendement vise à préciser les modalités d'information et de recueil de la signature du consommateur, à responsabiliser les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution et à conférer aux autorités de contrôle la capacité de s'assurer du plein respect des dispositions auxquelles ces acteurs sont soumis. Enfin, cet amendement tend à prévoir une obligation de conservation des enregistrements des appels de vente pendant une période de deux années. L'intention du Gouvernement est bien d'agir pour encadrer le démarchage téléphonique, pas la relation quotidienne entre assureurs et assurés ; les échanges liés à des contrats en cours ne sont pas concernés ni les échanges avec des clients professionnels. Ces dispositions s'appliquent en revanche aux nouveaux produits proposés à des particuliers. Le sous-amendement

L'amendement du Gouvernement vise à encadrer le démarchage téléphonique non sollicité réalisé par les distributeurs de produits d'assurances. Son objectif

eux confie le contrôle du respect des conditions d'honorabilité des courtiers à l'Orias, tant pour les dirigeants que pour les salariés. En cohérence avec cette disposition, il conviendrait de confier à ce même organisme l'ensemble du contrôle des conditions d'accès et d'exercice d'activités, ainsi que le respect des exigences professionnelles et organisationnelles. À ce jour, l'Orias exerce déjà une partie des missions prévues par la présente proposition de loi. Par conséquent, l'exercice par l'association professionnelle de la vérification des conditions d'accès d'exercice de l'activité des courtiers, ainsi que le respect des exigences professionnelles aboutirait à dédoubler les missions de l'Orias. Par ailleurs, je souligne que cela représenterait une charge administrative et financière non négligeable pour l'association professionnelle.

suivants du code des assurances. Pour l'ensemble de ces raisons et parce qu'il vaut toujours mieux faire simple que compliqué, je vous remercie d'apporter votre soutien à cet amendement. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, secrétaire d'État. La modification apportée par la commission sur ce point précis tend à réserver à l'Orias l'ensemble des vérifications d'honorabilité érigées par la loi, qu'il s'agisse de l'honorabilité des dirigeants ou de celle des salariés. La vérification de l'honorabilité des dirigeants est d'ores et déjà une compétence de l'Orias, et le Gouvernement n'entend pas y toucher. En revanche, nous avons la conviction que les associations peuvent aussi accompagner les entreprises de courtage pour les aider à remplir leurs obligations d'honorabilité. Par exemple, elles peuvent aider les dirigeants à collecter les déclarations de leurs salariés, comme le droit l'exige. Le Gouvernement propose donc de revenir au texte antérieur pour permettre cet accompagnement.

Mme Catherine Dumas. La proposition de rédaction du nouvel article L. 513-3 du code des assurances vise à mettre à la charge des associations professionnelles une obligation de vérification des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de ses membres, ainsi que de leur respect des exigences professionnelles. La rédaction actuelle de la dernière phrase de l'alinéa 4 tend à retenir une interprétation extensive de la notion d'exigence professionnelle, qui engloberait l'ensemble des exigences applicables à la profession, qu'elles soient d'origine législative ou réglementaire. Cela contreviendrait expressément aux dispositions des articles 12, 3 et 10 de la directive sur la distribution d'assurances (DDA), qui autorise les États européens à déléguer à des associations professionnelles le contrôle des conditions d'accès à la profession. La présente proposition de loi s'inscrit d'ailleurs dans cette démarche. Ces mêmes articles interdisent aussi de déléguer tout autre contrôle à des associations professionnelles et les réservent expressément et exclusivement aux autorités nationales compétentes. Aussi, pour lever toute ambiguïté, qui inscrirait potentiellement le présent texte en violation de la directive sur la distribution d'assurances, il est proposé de compléter l'alinéa comme suggéré afin de cantonner les exigences professionnelles aux seules conditions de capacité professionnelle et de formation continue. Il est également proposé de modifier l'alinéa 35 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement, ainsi qu'à leurs mandataires, dans les mêmes termes.

La commission s'est opposée au transfert de ces missions à cet organisme, constatant par ailleurs que ce registre n'est pas adapté pour les mettre en oeuvre. De plus, cet amendement aurait pour conséquence de priver les courtiers en assurances et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement d'une plus-value que nous percevons comme essentielle dans la proposition de loi, à savoir l'accès à un service de médiation.

l'inconvénient d'être une charge administrative supplémentaire pour les associations professionnelles, avec une fiabilité moins élevée, puisque celles-ci n'ont pas directement accès au casier judiciaire. Essayons de faire simple et efficace

ainsi que des codes homologués par le ministre chargé de l'économie. Toujours en matière de pratique de vente et de protection de la clientèle, le législateur a confié à l'ACPR la mission de veiller au respect des codes de conduite approuvés par elle, à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de la profession organisme constate ou recommande. Ainsi, il appartient réglementairement à l'ACPR, et à elle seule, de dégager des bonnes pratiques à l'intention des professionnels soumis à son contrôle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. Il vous est donc proposé de modifier l'alinéa 17 en ce sens. Quel est l'avis de la commission ?

à réduire les charges, notamment juridiques et financières, qui seraient supportées par les dirigeants des cabinets de courtage si la réforme était mise en oeuvre. Quant aux associations professionnelles chargées de cette mise en oeuvre, il est essentiel qu'elles aient le temps, avant même l'entrée en vigueur du dispositif, de s'organiser non seulement sur le plan matériel,

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons une modification de l'alinéa 116 pour substituer à la date du 1avril 2022 la date du 1 janvier 2023, soit neuf mois de délai supplémentaire pour une bonne intégration des nouveaux dispositifs de la réforme par les acteurs concernés. Catherine Dumas, pour présenter l'amendement n° 6. La proposition de loi alourdit les obligations des cabinets de courtage en mettant à leur charge une condition supplémentaire d'adhésion à une association professionnelle. La crise sanitaire liée à la pandémie s'est transformée en une crise sociale et économique qui affecte, à des degrés d'intensité variable, l'ensemble des secteurs d'activité. Elle se traduira immanquablement par une montée sensible du taux de chômage et une augmentation du nombre de défaillances d'entreprises. Alors que leurs chiffres d'affaires de 2020 ont été relativement préservés en raison des particularités de notre cycle de production, les courtiers vont entrer dans une crise à leur tour et y demeurer jusqu'à ce que leurs clients parviennent à se redresser. La mise en place de cette réforme, dans le contexte actuel, va venir accroître la pression juridique et économique sur les cabinets de courtage. Quant aux associations professionnelles qui sont chargées de mettre en oeuvre cette réforme, il est essentiel qu'elles aient le temps, avant même l'entrée en vigueur du dispositif, de s'organiser tant sur le plan plan matériel, notamment par la création d'un système informatique dédié qui, à ce jour, n'existe pas, que sur les plans humain et financier. Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement vise à préserver la pérennité du secteur de courtage, compte tenu du contexte actuel, et à laisser le temps aux différents acteurs de se préparer à une mise en application efficiente des mesures issues de cette réforme.

l'avis de la commission ?